Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Pas d'observation, le procès verbal est adoptée sous réserve d'usage. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à l'industrie verte dans la discussion des articles. Nous sommes parvenus à l'article 8. Et sur l'article 8, j'ai une prise de parole de monsieur le rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président. L'article 8 étant la liste des projets éligibles à la procédure de déclaration de projet. Cette dernière permet la mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme plus rapidement qu'avec les procédures classiques de révision ou de modification. Elle peut être à l'initiative de l'État ou à l'initiative des collectivités. Le texte initial du projet de loi visait les projets industriels je cite qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Ces secteurs seraient définies par décret en Conseil d'État. De nombreux au même moment, en commission comme en séance souhaité préciser les activités concernées. La commission des affaires économiques ne souhaite pas ouvrir cette boîte de Pandore pour 2 raisons. Premièrement en élaborant dans la loi une liste de secteurs fermé nous privons le pouvoir réglementaire de toute capacité d'adaptation face aux futures évolutions technologiques. Nous perdons ainsi nous perdrions ainsi beaucoup dans un agilité et donc pense potentiellement en temps ce qui serait exactement le contraire de ce à quoi vise le projet de loi. Deuxièmement, le bénéfice de la déclaration de projet ne se limite pas au secteur explicitement cités dans cet article. Toute opération d'aménagement d'intérêt général peut en bénéficier. Y compris toutes sortes d'implantation industrielle. Une liste fermée dans la loi pourrait être interprété comme exclusive d'autres secteurs, là aussi nous perdrions en agilité et on adaptabilité enfin tous les secteurs visés par les amendements sur lesquels nous aurons à nous prononcer sont compris dans le règlement dans le Industrie zéro Net actuellement en cours de négociation et comme nous l'a dit le ministre lui-même constituera la base minimale pour la liste qui sera élaboré par décret ainsi tous vos amendements sectoriels ont-ils vocation à être satisfait dans un avenir proche pour cette raison, il ne paraît pas souhaitable d'alourdir la loi.

L'esprit de ce projet de loi et de faciliter l'implantation et le développement des sites industriels en accélérant les délais mais au détriment, une fois encore, hélas, du droit de l'environnement et au détriment du débat public. Cet article 8 n'échappe pas à cela en accélérant le processus d'autorisation des nouveaux sites industriels afin de permettre aux différents projets d'un ce qui, d'industrialisation dites vertes d'aboutir plus rapidement. Ygéna réalise ainsi la déclaration de projet à plusieurs types d'industries dans des secteurs largement défini par décret le périmètre de cet article et ainsi on ne peut plus floue, et c'est ce que nous regrettons en particulier nous nous opposons fortement à ce dispositif, la déclaration de projet devrait être exceptionnelle et non un mode d'aménagement du territoire. Si avec la déclaration projet et les gains en termes d'accélération des implantations sont bien réels. La balance bénéfice-risque ne nous paraît pas équitable. C'est une planification descendante au lieu de demander au projet industriel de s'insérer dans le projet de territoire et ceci avec une élaboration collective on modifie ce dernier pour laisser les porteurs de projets, décider de leur implantation. Sans réel encadrement des potentiels nuisances et risques environnementaux qui peuvent accompagner toute activité de fabrication. Le Conseil d'État, s'interroge lui-même sur le cumul des cas où une modification des règles local d'urbanisme peut être imposée aux collectivités territoriales. Le dernier cas en date n'étant pas plus vieux que celui introduit par la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables qui avait toutefois le mérite de mieux cadrer le périmètre. Par ailleurs, nous pouvons douter de l'efficacité de cette mesure, la loi ASAP votée en 2020 avait déjà simplifier les démarches pour obtenir des autorisations administratives d'implantation d'usines sans effet vraiment visible sur la réindustrialisation. La commission a d'ailleurs largement élargi le Champ des bénéficiaires de la déclaration de projet ce qui aggrave la portée de cet article pour toutes ces raisons, nous proposons sa suppression. Avis de la commission. Merci monsieur le président. Chers collègues, l'inclusion des projets industriels verts dans le Champ des opérations qui peuvent bénéficier de la déclaration de projet répond. À un objectif d'affichage plutôt qu'il nous réellement de nouvelles possibilités. En effet, la déclaration de projet peut être mobilisés par l'État ou par les collectivités sur quasiment tout projet d'aménagement et la jurisprudence a régulièrement admis sa mobilisation pour des projets industriels, pour peu qu'ils représentent un caractère d'intérêt général et pas seulement comme vous le dites exceptionnelles. Il s'agit donc de surtout de faire ici valoir aux collectivités qu'elles peuvent utiliser cette procédure si elles en éprouvent le besoin pour des projets d'industrie verte sur le fond les gains réels puisque la durée moyenne de modification d'un PLU sans utiliser cette procédure de mise. La procédure de mise en compatibilité. Vous le savez, de 2 à 4 ans. Beaucoup trop pour un projet industriel. Je rappelle que lorsque c'est l'État qui prend la décision, il ne peut pas porter atteinte aux éléments essentiels de ces documents ce qui apporte des garanties aux collectivités. C'est pourquoi ce sera un avis défavorable. Si monsieur le président. Même avis. On n'oppose pas l'écologie lente à l'industrie rapide ou l'écologie inefficace à l'industrie efficace on doit être capable de faire de l'industrie. Qui non seulement respecte l'environnement, mais même concours à la lutte contre le réchauffement climatique et préserver l'environnement et je pense que c'est l'objet important de cet article que nous souhaitons évidemment préservée et c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à cet amendement de suppression. Le rapporteur a très bien présenté l'article mais pour vous donner une idée des avis que nous allons du coup si vous m'y autorisez. Monsieur le Président. Très rapidement pour la suite de l'examen. Nous souhaitons pouvoir préserver la capacité du gouvernement à listé par décret le rapporteur a très bien exprimé. Pourquoi les secteurs qui seront concernés. Tout ce qui sera fixé dans la loi permettra malheureusement d'éviter d'en rajouter ou en tout cas d'alourdir. De manière trop forte notre capacité collective à ajouter de nouveaux secteurs, Le caractère général de cet article, y compris monsieur le rapporteur pour la logistique. De manière à ce que le décret puisse préciser tout ça, les parlementaires seront évidemment associés à la rédaction du décret nous sommes défavorables à cet amendement de suppression et nous serons défavorables à l'ensemble des amendements qui visent à trop préciser donc trop encadrer la liste. Concernés. Merci. Merci je mets aux voix l'amendement cinq avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre.

Il nous faut des des biocarburants pour pour nos transports. C'était important pour l'avenir dans une perspective de de transition vers une économie plus verte et bien entendu la production de biocarburants doit servir à décarboner le secteur de la mobilité en général et plus particulièrement celui de de l'aérien. Donc encourager le déploiement des installations de production de biocarburants en France. Est un levier indispensable pour l'élaboration d'une industrie souveraine compétitive écologique. Le développement des biocarburants et donc la condition sine qua none pour aboutir à des résultats concrets en matière de décarbonation de nos transports et surtout pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est pour ces raisons qu'il convient de de les introduire ces ces biocarburants dans le Champ de l'article 8. Ce que propose cet amendement.

ou incluses dans le zéro le le 0 Act européen ou le justement cette libéralisation pour permettre une ouverture et la possibilité d'adapter justement notre réindustrialisation sur tous les projets de souveraineté comme industrie verte ce sera donc un avis défavorable.

Oui, monsieur le président, mes chers collègues, vous le savez, le processus de production de silicium et vital en fait pour la fabrication de cellules photovoltaïques. Il nécessite un apport en carbone sans aucune autre alternative et de ce fait utilise encore aujourd'hui une forte quantité de charbon fossiles. Or pour atteindre la neutralité climatique avec une demande croissante de silicium. L'approvisionnement de l'industrie européenne en bio-carbone issu d'une gestion durable des forêts doit augmenter pour se substituer au charbon fossiles. L'idée donc de d'intégrer ces installations de production du carbone dans la liste des projets d'intérêt national majeur, c'est le cas dans l'Aube du groupe solaire dont la technologie est mondialement reconnu. C'est l'objet de cet amendement.

monsieur le président. Excusez-moi je, je voulais dire que je le retire s'désir d'avoir la garantie de l'inclusion dans les décrets de la production de biocarburants, mais je souhaiterais l'entendre de la part du ministre. À

Oui, les technologies de décarbonation nécessite de plus en plus la construction d'usines de site de stockage et de logistique à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des matières premières et des et, des produits finis. Ces sites sont soumis aux mêmes règles, les difficultés que les usines. C'est pourquoi le présent amendement propose d'étendre les dispositions de l'article 8 aux installations de stockage des produits ou équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorable au développement durable.

Merci monsieur le président. Les 2 amendement vise à prendre en compte les infrastructures logistiques, liés au processus de production pour les activités visées par l'article. L'amendement 61 restreint cette facilité aux infrastructures logistiques directement liées au processus de fabrication et d'assemblage des chaînes de valeur dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. L'amendement 358, quant à lui est plus imprécis puisqu'il ne pourrait il ouvrirait plus largement la porte. Y compris Monsieur le ministre à des types d'entrepôts logistiques que nous n'avons pas forcément envie de favoriser et qui ne participent pas au processus de création. Je demanderai donc le retrait de l'amendement 358 au profit du 61 à défaut ça sera un avis défavorable pour le 358 est favorable pour le 61. D'accord avec le gouvernement. Non même avis en précisant que je serais sans doute défavorable pour autant 61 donc faut que tout le monde soit conscient de l'avis du gouvernement sur ces deux amendements qui il est vrai, sont liées. C'est-à-dire que le gouvernement est défavorable sur les deux en toute. Non c'est pas ce que j'ai. Beaucoup de monsieur le président. Pas de problème. Le 358 Madame Paoli-Gagin retirer donc je mais ou vois le 61 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement. Qui est pour.

Merci Monsieur le Président l'amendement me semble contre-productif dans la mesure où il restreint le dispositif uniquement aux petites et moyennes entreprises au détriment des installations plus important tout aussi légitime en bénéficier. Je vous signale, chers collègues, en précisant que les activités participant indirectement aux chaînes de valeur des secteurs favorables au développement durable qui peut qui pouvaient bénéficier de la déclaration de projet. La commission des affaires économiques viser précisément le cas de ses sous-traitants dont l'installation rapide peut être en effet crucial pour les industries de 1er rang visés à l'origine par l'article, votre demande ne semble donc satisfaite, ça serait une demande de retrait ou un avis défavorable.

Avec les secteurs favorables au développement durable. Là j'ai peur qu'on ouvre, non seulement la boîte de Pandore. Mais je dirais la foire à la saucisse là tout sera possible Lewis qui rentrerait éventuellement dans la fabrication d'un bâtiment qui lui même. Abriteraient des éoliennes, des pompes qui permettraient de fabriquer des tuyaux qui eux-mêmes permettrait éventuellement de transformer de transporter le CCAS, le verre qui pourraient entrer dans des panneaux solaires mais aussi dans des vitres de bâtiments donc on on souhaite plutôt. se cantonner et se contenter des des activités directement liées au secteur favorable au développement durable et donc défaveur pardon on restaure. Du coup, la rédaction initiale modifié dans le sens de l'indirect par la commission. Avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre de la commission a jugé utile de préciser que dans certains cas les installations concourant indirectement aux chaînes de valeur pourront aussi être éligible. Il pourrait par exemple s'agir de certains sous-traitants ou de certaines activités de services nécessaires à ces industries de 1er rang. dates Atlas à des Data centers, des choses comme celles-là et qui pourrait avoir besoin de bénéficier des mêmes facilités pour s'installer rapidement sur le territoire au risque de mettre en péril le projet initial. Je rappelle qu'en aucun cas la mention de ces types de projets à l'article L. 306 du code de l'urbanisme ne fait obligation de recourir à la déclaration de projet, un projet ne peut se faire l'objet de déclarations de projets que s'il répond à un critère d'intérêt général. Les collectivités ou l'État lorsqu'il s'agit de lui auront le discernement suffisant pour décider s'il est ou non pertinent et justifié de recourir à cette procédure au cas par cas, ce sera donc un avis défavorable. Interrogatif sur cette volonté d'élargir. À l'ensemble de tout ce qui pourrait concourir on pourrait et peut-être qu'on devrait dans cette logique pousser plus loin et et veiller à ce que les équipements hôteliers susceptibles d'accueillir d'accueillir les personnels concernés, à ce que la restauration, les lieux de loisirs, les lieux de culte puissent aussi bénéficier je pense qu'à un moment donné il faut limiter ces procédures exceptionnelles au strict nécessaire et que cette idée de toujours élargir et de déroger aux règles et au fond une remise en cause permanente des droits de l'environnement et des droits de l'urbanisme et ça n'est pas acceptable. Merci je mais on voit le 314 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Le 38 Madame Paoli-Gagin. Oui, monsieur le président, la rédaction actuelle de cet alinéa vise uniquement les technologies favorables au développement durable. Cela risque d'exclure des activités relevant des secteurs traditionnels qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, les activités de maintenance réparation réemploi rétro feat remanie factura de biens d'équipements tels que les machines industrielles risque de ne pas répondre à la définition de la technologie en faveur du développement durable, je précise que je suis prête à retirer cet amendement si j'ai un engagement Express sur la garantie. Décréta les réglementaire de la part du ministre. Monsieur le président, cher collègue, votre amendement sera satisfait puisque la décarbonation de l'industrie et précisément l'un des principaux objectifs de ce projet de loi industrie verte. Je ne vois pas comment les secteurs qui sont favorables au développement durable. Visé par cet article pourrait ne pas comprendre les activités contribuer contribuant pardon à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone que vous citez, ce sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable. le secteur l'atteinte des objectifs de neutralité carbone est un peu trop large pour que je puisse m'engager au banc de manière explicite et systématique à ce que tous les secteurs y soient intégrés, mais en tout cas telle que rédigée. Par votre amendement. Il me semble évident que les secteurs que vous avez en tête, nous devrions les avoir aussi en tête, donc je suggère le régime.

En plus des technologies favorables au développement durable listés par décret les industries participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des énergies renouvelables, ainsi que l'hydrogène renouvelable. Les opportunités d'industrialisation de tous les secteurs d'énergies renouvelables sont en effet nombreuses dans la mesure où les filières industrielles d'excellence sont déjà ancré sur le territoire. À l'image de l'éolien en mer. 4 des 12 sites industriels stratégiques qui existe en Europe sont situés en France, c'est ce que une chaîne de valeur complète soutenu par un écosystème portuaire performant. Par ailleurs, certaines filières sont moins visibles dans le débat public et présente pourtant de très important potentiel d'industrialisation à l'image par exemple la filière de production de combustible bois haute performance de la filière de la petite hydroélectricité qui contient un tissu important et dynamique de PME en particulier dans le domaine électromécanique. Ainsi qu'elle fait. De la filière des énergies de récupération en particulier associé à la valorisation énergétique des déchets qui possède encore un potentiel important pour contribuer à la décarbonation des territoires et des industries s'agissant encore des énergies marines renouvelables. On peut noter que les turbines construites par les industriels français bénéficie d'un très fort contenu local. Le texte gagnera ainsi un quartier sera d'autant plus sécurisant. Si toutes les énergies renouvelables sont cités précisé dans la rédaction, ce qui permettra de lever toute ambiguïté sur le chef de l'application de l'article 8. Monsieur le président. Chers collègues, pour les mêmes raisons que précédemment, je demande le retrait de cet amendement ou à des fois un avis défavorable puisqu'il vise l'hydrogène ainsi que les secteurs des énergies renouvelables, éolien, solaire, géothermie biogaz. Je n'imagine pas un seul instant que votre amendement ne soient pas satisfaits.

public. Madame Billon. Merci Monsieur le Président. Cet amendement déposé par nos collègues. Anne-Catherine Loisier qui visent à à n'exclure aucune solution favorable au développement durable, des mesures de simplification de procédure prévue pour les industries vertes. Aujourd'hui, le qualificatif technologie est trop restrictif et ne permet pas d'inclure des filières de production de matériaux durables et bio-sourcés comme le bois pour autant l'industrie du bois participe au travers des différents usages qui sont faites de ce matériau stockage du carbone biochimiques aussi le développement de ces filières de matériaux durables est nécessaire pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050. C'est le sens de cet amendement. Merci. Merci le de 362 identique. Madame Beujin. Oui, monsieur le président. Il est il est défendu mais là encore, nous avons besoin de garanties. Commission. Oui, monsieur le président, chers collègues. Donc pour ces deux amendements de 135 362 je vous rejoins sur le fait que le développement durable c'est pas seulement de l'innovation et des technologies de rupture bien sur le bois est un et Martin. Un matériel un matériau merveilleux à de multiples égards pour contribuer au développement durable parce que ils stockent du carbone. Pour autant, je vous invite à lire Le Courrier Picard d'aujourd'hui qui signale que les forêts françaises ne ne ne ne ne remplissent pas complètement, je dirais, cette fonction est pas autant en tout cas qu'il était prévu. Peut-on pour autant considérer que l'ensemble justement de la filière bois est favorable au développement durable. Qu'une scierie où une fabrication de meubles à l'autre bout de la France. Participe à prendre le virage de la transition écologique la taxonomie européenne prévoit par exemple de favoriser les activités visant à gérer les forêts de façon durable ce qui est déjà plus restrictif. La mention matériaux semblent vraiment trop large, car elle ne fait pas la distinction entre entre les usages, ce sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable. telle qu'il rédigé l'amendement, il est un peu trop large avec des notamment pour nous permettre, nous nous autorise à y être favorable mais dans le décret. Je m'y engage le bois et la filière bois ils sont clé et ils seront bien intégré au décret en question donc retrait.

Cet amendement déposé par notre collègue Claude Kern. Le, l'article 8 du projet de loi sincère au sein du chapitre 5 visant à faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes en leur Current cet article 8 prévoit de compléter les dispositions de l'article L. 300 tiret 6 du code de l'urbanisme, lequel prévoit pour les projets. Pour lesquels l'État et les et ces établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements prononce par une déclaration de projet le caractère d'intérêt général. Celle-ci emporte mise en compatibilité accélérer et simplifier les documents d'urbanisme, donc c'est l'objet de de cet amendement et donc. Je vous laisse répondre. Merci. Enfin pas moi un. Avis de la commission. Monsieur le président. Chers collègues effectivement je ne suis pas favorable à cet amendement car il touche au verdissement des usages. Et non spécifiquement au verdissement de l'industrie tout bien considéré, une usine de recyclage peut être très peu décarboné. Et donc, assez peu favorable au développement durable. J'ai, si j'ai par exemple elle fait une consommation excessive d'énergie. Non non non décarboné pour fonctionner. Donc je rappelle en revanche que l'article 306 du code de l'urbanisme ne fait aucun obstacle à ce qu'une collectivité mobilise la procédure de déclaration de projet au profit d'une usine de recyclage. Si celle-ci peut être considéré comme d'intérêt général dans son périmètre. Ce sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Gouvernement de ma vie. Alain Billon retirer merci. 3 amendements en discussion commune. Ben justement Madame Billon, vous faites les 113 et 114. Alors merci monsieur le président. Ces deux amendements. Alors l'article 8 du projet de loi relatif à l'industrie verte c'est ce ce ce texte évidemment prévoit pour que les pouvoirs publics locaux et nationaux puissent se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général de certaines installations industrielles et sont notamment visés les installations industrielles industrielles de fabrication ou d'assemblage mais aussi les installations R&D ou d'expérimentation des produits et équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs de technologie favorable au développement durable. Le présent amendement et donc le 113 rectifié vise donc à clarifier la portée de l'article 8, en précisant que les technologies favorables au développement durable mentionnés dans l'article incluent notamment les technologies de capture de transport de séquestration ou d'élimination de carbone. l'amendement 114 rectifier toujours déposé par notre collègue Claude Kern. Ce, cet amendement vise donc à clarifier la portée de l'article 8, afin de faciliter l'implantation des dispositifs de capture de transport de séquestration ou d'élimination de carbone. Voilà monsieur le président. en mentionnant l'implantation des dispositifs de capture de transport de séquestration d'élimination du carbone, nous le savons, l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère due aux activités humaines est la cause principale du réchauffement climatique. C'est pourquoi les différentes méthodes permettant de retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère et de le stocker durablement ont un rôle primordial primordial à jouer dans les années à venir. L'élimination du carbone atmosphérique de se développer dans un cadre législatif clair et stable. Je vous remercie. Merci. Il y avait de la commission sur les trois amendements. Monsieur le rapporteur. Prendre l'argument de la liste à la Prévert qui vaut également pour les amendements 113 114 et 117. Comme les biocarburants. Les technologies sont bien incluses dans la proposition du règlement industrie zéro Net votre demande sera donc in fine est satisfaite, ça sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable.

du carbone fatale en tout cas pendant longtemps et donc on a besoin de mettre paquet là-dessus ne l'incluant pas dans la loi puisqu'on va le faire dans le décret. Mais je m'y engage devant le Sénat. Que retrait des favoris. Audrey. Merci. Je passe au 50 Madame Paoli-Gagin. Oui, monsieur le président, on le sait dans le contexte d'épuisement des ressources. Le recours aux matières premières. Du recyclage va jouer un poids de plus en plus important, notamment pour nous fournir du lithium. Du cuivre recyclé pour les batteries des véhicules électriques mais également des aciers recyclés moins émetteurs de CO2 que l'acier issus de minerai de fer le présent amendement propose donc de reconnaître les projets d'installations de recyclage comme des projets d'industrie verte afin d'encourager leur réalisation et concilier l'ensemble des efforts qui doivent être menées en matière de transition écologique et de réindustrialisation de la France, là encore. Retrait versus garantie. Merci commission. Monsieur le président. Chers collègues, sans vouloir réouvrir le débat que nous avons très intéressant que nous avons eu hier votre amendement effectivement est intéressant car il considère le recyclage. Non, en soi, mais en tant qu'il permet de fournir des intrants. Pour l'industrie sans piller les ressources naturelles. Cette réflexion manque effectivement dans le projet de loi, nous l'avons signalé hier, qui considère le verdissement de l'industrie que sous le prix le prisme pardon de la décarbonation. Recycler les matières premières critiques nous rend aussi moins dépendants de nos fournisseurs étrangers. C'est aussi un pas de plus vers la souveraineté nationale. Dans le même temps, je ne suis pas favorable à alourdir le texte, ce sera donc un avis de sagesse. Après l'avis du gouvernement. Le 378 n'ait pas défendu le 351 madame Paoli-Gagin.

Et défendu avis de la commission sur le trois. C'est la liste à la Prévert comme tout à l'heure, ça sera donc un avis défavorable. Ouais. Retrait ou défavorable pour les mêmes raisons. Il est. Il est retiré. Voilà je mets aux voix l'article 8. Oui Monsieur Salmon. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, avec cette liste d'amendements, nous voyons bien que, hé bien nous sommes train d'ouvrir. Très large autour de ce qui peut concerner l'industrie verte et on a bien ciblée dès le début. Cet cet écueil en disant, que hé bien il ne faut pas brader aujourd'hui les droits de l'environnement, les droits de l'urbanisme et la consultation du public ça s'impose, il faut une appropriation de cette industrie verte de cette industrie nécessaires à la transition écologique mais cela ne doit pas se faire au détriment de ses consultations et de l'intégration des collectivités territoriales dans la décision. c'est pour ça que nous avions proposé la suppression de certes article parce que même si nous sommes pleinement favorable à la réindustrialisation et la relocalisation. La définition de l'industrie verte, on l'a déjà dit à plusieurs moments n'est pas présente clairement dans cette. Dans ce projet de loi. Merci. Merci je mets aux voix l'article 8 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté après l'article 8, le 352 madame Paoli-Gagin. Merci monsieur le président, le Silicium, on l'a déjà vu c'est un matériau critique et il est considéré comme telle par le règlement européen. Il est indispensable à la fabrication des cellules de panneaux photovoltaïques des batteries, des micro-, puces et des matériaux de haute performance. Aujourd'hui, nous le savons, la Chine domine. La chaîne d'approvisionnement mondiale de ce matériau critique et les émissions moyennes de CO2 de la production de silicium sont passés de 8 tonnes. En 95 à 11 tonnes en 2019. 1er producteur européen de silicium. La France bénéficie d'un écosystème pionnier dans le domaine du carbone renouvelable. Comme alternative au charbon fossiles. Nous avons ainsi l'occasion unique de développer la première industrie du Silicium véritablement verte au monde d'où la demande de publication. Par le gouvernement d'un rapport sur le verdissement de notre industrie du Silicium dans une logique de recyclage d'économie circulaire comme on l'a évoqué tout à l'heure. S'il avait de la commission, c'est le rapporteur. Si effectivement l'approvisionnement en matériaux critiques étaient est important pour le verdissement de notre. De notre industrie il ne me paraît pas de bonne politique de demander un rapport au Parlement sur chacun des intrants. Même si hier j'ai précisé que la règle générale. par ces exceptions ça sera quand même je dirais la la jurisprudence du Sénat qui va. S'appliquer aujourd'hui et ce sera donc un avis défavorable. Je ne veux pas dire qu'il est satisfait, mais je pense qu'il y a suffisamment d'informations en tout cas pour éviter un nouveau rapport retrait ou des favoris. Retrait. Ah il est retiré. Ça. À l'article 9. Monsieur le rapporteur. Une prise de parole. Oui, merci monsieur le président. Mes chers collègues, l'article 9 crée une nouvelle procédure accélérée de mise en compatibilité des documents de planifications et des documents d'urbanisme pour les projets dits d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, vous le savez, les associations d'élus ont exprimé leurs plus vives réticences à l'égard de cet article qui après la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Après la loi sur l'accélération du nucléaire, mais un nouveau coup de canif dans les compétences d'urbanisme du maire et bafoue le principe de subsidiarité qui devrait pourtant toujours guidé la répartition des compétences dans le cadre de la décentralisation. Pour la commission aussi l'intervention unilatérale de l'État dans les documents de planification et d'urbanisme est une ligne rouge il y a d'ailleurs une incohérence à donner aux régions une compétence de planification industrielle à l'article 1er et à leur refuser tout rôle pour les grands projets à l'article 9. Cependant, la commission a aussi été sensible à l'objectif d'accélérer les implantations des très gros projets industriels qui peuvent représenter des milliards d'euros d'investissements des milliers d'emplois. En outre, vu le cahier des charges. Le nombre de projets concernés chaque année devrait se comptaient sur les doigts d'une seule main. C'est pourquoi la commission n'a pas souhaité supprimer purement et simplement cet article mais l'a profondément remanié pour garantir la participation effective des collectivités à toutes les étapes de la procédure. Premièrement, pour sortir de la logique jacobine et purement descendante promue par le gouvernement. Nous avons permis aux régions en lien avec les collectivités, les collectivités locales, pardon de faire reconnaître elles aussi des projets industriels, d'intérêt national majeur alors que le texte initial réserver cette cette possibilité à l'exécutif. Deuxièmement, nous avons prévu une phase de dialogue d'un mois entre l'État et les collectivités avant. Engagement de la mise en compatibilité est conditionné cette dernière à l'accord des collectivités concernées. Le gouvernement vous dira certainement que notre système est compliqué et chronophage. Nous lui répondrons que l'acceptation locale est essentielle au succès du déploiement d'implantation d'industries vertes dans les territoires. Il serait contreproductif de limiter la concertation avec les élus et avec les habitants pour accélérer les projets. C'est ainsi que naissent les notre dame des Landes et autres. Monsieur lui. Votre fan club monsieur le rapporteur. Monsieur Buy. Merci monsieur le président, mes chers collègues, quelques mots sur cet article car nous considérons la nouvelle procédure instaurée par l'article 9 comme parfaitement justifiée. Étant donné l'importance des projets concernés qui se chiffrent en milliards d'euros mais également eu égard à la concurrence internationale féroce qui est l'oeuvre concernant les implantations des grands sites industriels. a annoncé lundi un accord avec l'entreprise untel pour l'installation à Magdeburg d'une méga Fab à 30 milliards d'euros pour laquelle l'Allemagne versera une aide de 10 milliards d'euros, un euro d'argent public donc pour 2 euros d'argent privé cette annonce démontre s'il en était nécessaire que nous devons prendre des mesures drastiques. Si nous voulons implanter chez nous des activités industrielles du futur et ne pas rater le wagon de l'industrie l'industrie du XXIe siècle. L'article 9 est une partie de réponse à cela car en plus d'accélérer les procédures, il offre une stabilité une prévisibilité aux porteurs de projets 2 éléments fondamentaux pour des entreprises industrielles. L'esprit de cet article n'est pas de passer au-dessus des élus mais bien de renforcer l'attractivité de nos territoires pour attirer des implantations d'activités industrielles. Nous sommes attentifs à ce que les implantations ne se fasse pas contre contre les élus. C'est pourquoi nous proposerons d'instaurer un recueil de l'accord du maire ou du président de l'EPCI concerné par l'implantation préalablement à l'engagement de la procédure ici instauré nous présenterons également un amendement revenant sur le dispositif permettant aux régions d'Esquire de droit des projets dans la liste des projets d'intérêts nationaux majeurs introduit en commission. Monsieur le rapporteur. Loin de nous l'idée de vouloir poser des difficultés, mais il semble important que le Sénat veillent à préserver l'équilibre de la répartition des compétences, les régions, tout à fait la possibilité d'être à l'initiative, nous les encourageons mais nous pensons nécessaire d'établir une limite claire l'intérêt national n'est pas déterminé par les régions. Nous y reviendrons dans la discussion de nos amendements. Merci. J'ai trois amendements en discussion commune que s'ils sont identiques, je précise tout de suite que ces amendements de suppression vont faire l'objet d'un scrutin public. À la demande du groupe écologiste, donc merci de vous y préparer le 142 Monsieur Salmon. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre sur le rapporteur ma chère collègue. La commission a fort heureusement modifié cette Arctique particulièrement problématique à savoir soustraire à la compétence du droit commun des collectivités les autorisations d'urbanisme concernant des projets d'intérêt national majeur. Et ce, en vue de confier à l'État la décision de leur implantation. Cette mesure constituait une nouvelle et grave atteinte à la libre administration des collectivités pourtant concernés au 1er chef et en particulier leurs compétences local d'urbanisme. Cet article constituait lave de d'une méconnaissance de la part du gouvernement de la réalité des dynamiques industrielles territoriale et des conditions d'implantation réussie sans le territoire ça ne sera pas réussi mais cet article continue de poser un certain nombre de problèmes et met à mal le principe de non-régression du droit de l'environnement. Il vise là aussi à réduire les délais afférents aux autorisations d'urbanisme et vient d'ailleurs en complément des dispositions des articles 2 et 3 qui réduit se afférents. La procédure d'autorisation environnementale et réorganise les modalités de consultation du public, cela ne nous paraît pas acceptable d'autant que le texte étend le bénéfice de l'accélération à l'ensemble de la chaîne de valeur, avec un renvoie à une définition réglementaire de ce secteur. Concernés qui permettrait davantage d'adaptabilité et d'agilité, attention à ces 2 mots en l'absence d'encadrement. Nous ne pouvons souscrire à cette mesure. Je rappelle que pour les projets d'ENR les activités étaient bien lister. De plus, la Commission a prévu que les projets qualifiés d'intérêt national majeur puisse bénéficier d'une présomption de reconnaissance d'un impératif d'intérêt public majeur R 2 IPM pour que soient délivrer une dérogation à l'obligation stricte de protection de certaines espèces. Le Conseil d'État estime pourtant qu'il faut encore atterri cette reconnaissance automatique par des critères pertinents.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Même revu. Par la Commission comme il l'a été le rapporteur là l'expliqué l'article 9, mettent en place une nouvelle procédure dérogatoire de mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme et d'urbanisme locaux pour des projets d'intérêt national majeur qui répondent donc un enjeu de souveraineté national ou de transition écologique et ces projets seront décidées par l'État dans le cadre d'un décret. Le Conseil national d'évaluation des normes a émis un avis défavorable sur cet article. Considérant que l'implantation d'industries, d'intérêt national ne peut justifier qu'il soit dérogé à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales pour la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les associations, des représentants d'élus sont également opposés à l'article 9. Ce qu'il porte atteinte au pouvoir des maires et plus précisément aux compétences local d'urbanisme. Il transfère cet article la compétence à l'état pour délivrer les permis de construire et place le préfet comme interface unique du porteur de projet. Ce texte organise clairement l'ingérence de l'État dans les compétences des collectivités territoriales en matière d'aménagement du territoire. Monsieur le Ministre, nous avons besoin d'une clarification de la part du du du gouvernement. Comment peut-on afficher l'ambition de territorialiser davantage la politique industrielle de faire travailler ensemble, l'État et les et les collectivités d'organiser la planification industrielle à l'échelle des territoires. Ce qui suppose une concertation d'ampleur et à la fois prévoir que l'État pourra in fine et reprend dans la main sans concertation des élus locaux. Voilà. Pour toutes ces raisons. Notre groupe propose également la suppression de cet article 9. Merci le 274 monsieur. merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi je pense qu'il nous faut un débat qui dépasse largement. Ce seul texte et ce seul amendement d'ailleurs, je vous remercie. Sur le rapporteur de l'avoir essayé de trouver un point d'équilibre mais je pense qu'il nous faut un débat sur qu'est-ce qu'on a en même temps par intérêt national majeur. Et ensuite qu'on se donne une règle claire. Pourquoi ça fait déjà 3 textes hein sur l'implantation des énergies renouvelables de sur la question du nucléaire et maintenant le 3ème sur la réindustrialisation et à chaque fois, et je nous mets dedans donc c'est pas une critique envers untel ou untel suivant notre sensibilité. On dit on veut donner la main à l'État et il faut qu'il passe au dessus des collectivités et si on a une autre sensibilité non non les collectivités avant tout et même certains ont envisagé des droit de véto sur certaines plantations et donc je le dis, on ne peut pas avoir nous toutes et tous. Quelque chose à géométrie variable. C'est pour ça que j'entends qu'on ait un débat sur sur qu'est-ce qu'on considère d'intérêt national majeur et moi je considère que la réindustrialisation du pays, c'est l'intérêt national majeur. Les et le développement des énergies avec un grand service public et un monopole public pas comme vous l'entendez. Monsieur le Ministre, je pense que c'est un intérêt public majeur. Mais après on nous on une est clair. Soit on décide que l'État à la main sur tout. Et donc ah bah les collectivités ou alors on considère. Que à un moment donné. Le pouvoir des collectivités, des maires et des policiers municipaux doit donner leur avis ou est-ce qu'ils doivent même décisionnaires. Moi je pense qu'il nous faut trouver un point d'équilibre. Et que ça l'intérêt plus national majeur ne peut pas se faire sans les élus locaux et la population. Parce qu'autrement un certains nombres de projets sont vouées à l'échec. Et il n'y a pas. Sans les élus locaux et la population d'implantation réussie, quel que soit, que ça soit en matière énergétique ou amateurs industriel donc. Nous, on propose même s'il a une réécriture de de de d'abroger ce texte mais je vous le dis, Monsieur le Ministre. Il nous faut un débat d'ampleur sur l'intérêt national majeur. Merci monsieur le président. On est sur un sujet extrêmement important, et donc ces amendements de suppression me permettent de vous donner l'avis du gouvernement sur cette procédure que nous avons envisagé. Intégré dans le cas de ce projet de loi et que nous sommes évidemment prêts à faire évoluer à l'occasion des débats parlementaires. On parle ici de quelques projets. On parle ici de un 2 ou 3 projets par an qui au fond engage notre nation industrielle. Dans la compétition mondiale. La plupart des projets dont on parle depuis maintenant quelques heures quelques heures Allez du type championnat de France, championnat d'Europe, on est là pour aligner l'équipe de France, chacun a ses responsabilités extrêmement bien. Et la pratique que moi, j'observe tous les jours c'est qu'en général l'industrie française n'a pas de couleur de maillot. L'état, la région, le département les EPCI les communes sont toutes alignées pour développer, vous l'avez dit, monsieur le sénateur gay l'industrie dans le territoire. Là on parle d'un ou deux projets par an qui nous font passer dans la Ligue mondiale, pour lesquels on est en compétition avec le monde entier pour lequel chaque détail compte. Et pour lequel nous considérons en effet. Que sur ces cas particuliers. Nous devons pouvoir donner de la visibilité aux investisseurs internationaux et leur donner un interlocuteur unique. Et c'est la raison pour laquelle. Pour ses projets qui sont des projets de souveraineté qui sont des projets d'accélération majeure de la réindustrialisation et des projets d'accélération majeur de la décarbonation nous avons suggéré une procédure et ça a été dit sur lequel le Conseil national d'évaluation des normes avait un certain nombre de réserves et je le répète, nous sommes prêts à évoluer sur ce point. Nous avons considéré que l'État devait je dirais. Avoir le dernier mot et surtout la signature sur le permis de construire. Pourquoi, pour qu'on puisse dire. Aux investisseurs qui viennent nous voir, sur ces projets. La personne qui va s'occuper de vous, de A à Z, c'est monsieur le préfet, c'est monsieur Untel ou c'est madame untel. Vous souhaitez et c'est normal. Nous devons trouver une rédaction qui nous permet de le faire qu'évidemment les élus locaux puissent s'opposer à ce type de décision s'il considère que ce projet d'intérêt national n'a rien à voir chez eux. Et je vais vous dire une chose. Quelles que soient les dispositions qu'on serait prête à adopter aujourd'hui si on a un maire, ou un président de PCI qui est vent debout face à un projet. Je pense qu'on aura du mal à le mettre en oeuvre et on aura du mal à convaincre l'investisseur international en question. Que c'est là qu'il faut le mettre. Donc on est juste en train d'essayer de trouver dans le cadre de cet article. Une rédaction qui va nous permettre de vous rassurer sur fait qu'évidemment le maire ou le président de l'OPC, il pourra s'opposer à un projet qu'ils jugent inutile ou contre-productif pour son territoire tout en saturant tout en s'assurant pardon que la procédure soit visible transparence efficace pour celles et ceux qui souhaitent choisir la France dans la compétition mondiale. Dans le cas des échanges avec l'Association des maires de France. Je pense qu'une rédaction de l'article a été suggéré. Je pense que c'était par le sénateur Buy en commission, je pense qu'elle est à nouveau proposée dans le cas de l'examen de ce texte en séance, 293 si je ne m'abuse, sur lequel nous souhaitons donner un avis favorable. Je m'y engage d'avance. Monsieur le Président pour bien éclairer les débats de l'ensemble de cet article. Qu'est ce qu'il dit finalement, cet amendement. C'est dès le départ. Stop ou encore le maire ou le président de l'. Il peut dire, Stop ou encore. c'est la main. De l'élu local qui va permettre de dire dès le début. On y va, on se met sur l'autoroute, on avance tous ensemble et on gagne ensemble ou pas. Et à partir du moment que le maire ou le président de la piscine, nous aurons dit Banco, on y va, on se met dans une logique où effectivement là, le préfet, l'État prend la main pour s'assurer que l'interlocuteur unique puisse être aussi efficace que possible. C'est la rédaction à laquelle nous serons favorables. Le risque évidemment de celles que vous avez adopté en commission. Ben c'est que. Stop ou encore. En fait on ne sait pas bien, on verra plus tard, le maire finalement à la fin, pourra décider. Avec un risque que l'investisseur disent, dans ces cas-là ben vous êtes gentil mais je vais voir ailleurs. Voilà donc je pense que c'est vraiment un enjeu de modalités qui nous oppose plutôt qu'un enjeu de principe, nous sommes pour évidemment. Le mot final mais plutôt au début des territoires sur ses grands projets d'intérêt national, alignant l'équipe de France de l'industrie pour gagner la compétition mondiale. Je pense que la rédaction proposée par le sénateur lui permet d'y arriver donc espérons qu'on y arrivera aussi avis défavorable évidemment sur ces amendements de suppression.

un peu partout mais il a raison, il faut, il faut de la cohérence sur ces bancs et nous nous essayons dans notre groupe d'avoir c'est cette cohérence en n'ayant jamais le souci de brader les collectivités territoriales. Par contre dans la loi, accélération des énergies renouvelables. Nous avons été cohérent pour nous l'échelon le plus pertinent et légion l'échelon régional, puisque c'est par le biais d'estrade être que les régions ont la compétence économique et donc nous essayons toujours de nous caler là-dessus. Nous nous sommes opposés bien entendu à des véto des vetos qui n'avait aucun sens des véto. Sur la co-visibilité des véto sur. Les bottes en lien avec les ABF et les bâtiments historiques. il y a des moments il faut rechercher la cohérence et la cohérence ne peut se faire qu'avec les collectivités territoriales territoriale et avec l'appropriation. Par nos concitoyens de la nécessité d'avoir une industrie avec le moins d'impact possible une industrie vraiment durable et aujourd'hui. Nous sommes dans ces dans ces divergences dans ces dans ces moments de tension. Il faut essayer de ne pas les alimenter justement avec des projets qui tombent comme ça là. Du haut, il faut vraiment qu'on ait cette rencontre entre les collectivités territoriales et la planification nationale et c'est un enjeu décisif pour les années à venir.

ça y est, mission accomplie. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe et vous le savez parfaitement bien Monsieur le Ministre. Il faut parfois construire des logements pour loger des salariés, il faut parfois développer des instruments infrastructures ou des services publics de transport, il faut souvent. Accueillir des médecins dans des territoires qui sont de plus en plus des déserts médicaux et ce genre de chose parce que effectivement on parle à de grands projets. Qui nécessitent il faut parfois former les salariés qui n'ont pas forcément le niveau de formation requis pour les emplois proposés. Et donc et il faut travailler à l'acceptation. De ces projets et des éventuels désagréments que ça peut apporter aux habitants bien tout ça c'est le coeur de métier des collectivités et donc il s'agit pas pour leur faire plaisir, de leur donner un pouvoir, il s'agit de travailler ensemble à cette réindustrialisation et je. Quand vous dites Stop ou encore. Les collectivités ne demande pas à dire j'en veux, j'en veux pas. Elle demande à pouvoir participer à créer les conditions. Pour que des projets industriels. Qui peuvent renforcer et. Répondre aux problèmes de souveraineté de la France, créer des emplois. Reconquérir un certain nombre de secteurs stratégiques. Les collectivités peuvent veulent pouvoir créer les conditions au nom des habitants qu'elle représente pour accueillir ces entreprises et c'est en ça que nous saluons effectivement le travail qui a été faire fait par la commission et je pense notamment au fait que les collectivités elles-mêmes puissent faire reconnaître des projets industriels dans dans les grands projets nationaux d'intérêt stratégique mais qu'il nous semble qu'il faut aller plus loin dans le partenariat a créé entre collectivités, État et en fait toute la communauté nationale pour pouvoir accueillir des projets que l'on souhaite. Merci cher collègue. Donc je suis saisi du de monsieur Montaugé. Oui merci. Merci Monsieur le le président, Monsieur le Ministre, que j'ai j'ai pas eu franchement de réponse à à la question que j'ai, que j'ai posée c'est pas grave je je voudrais redire ce que j'ai dit en discussion générale. Notre société la nation française. A besoin d'un grand récit. Par rapport au monde émergents. Dont nous aurons. Besoin pour vivre. Correctement ensemble demain. Voilà et dans dans ce grand récit. Il y a effectivement. Et ses centrales. La question de l'économie dont nous avons besoin. Je pense que ce ce ce grand récit. Il faut le il faut le construire. Aujourd'hui il est distillée par bribes. Voilà, chacun ayant à reconstituer le le puzzle pour comprendre. Où on veut aller où on peut aller. Et dans ce dans Je le répète après ce qu'ont dit mes mes camarades. Mes collègues. Les collectivités locales, les maires, les présidents d'EPCI. Constituent des relais de sens. Des relais de sens pour faire comprendre et faire accepter notamment ses grands projets. Le texte qui nous est proposé ne me celui de la, de la, de la commission. Les places à une situation extrêmement difficile qui à quoi veut-on arrivé on veut arriver à gagner du temps à à monter ces projets rapidement. Moi moi je crains que si on ne on dessaisi de cette manière-là. Les élus locaux. On on va, on, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire des blocages comme on en connaît trop souvent. Pour des motifs dits divers et je pense que tout le monde comprend quoi je fais allusion. Voilà il faut il faut impliquer d'emblée telles que la loi le permet aujourd'hui, sans rien changer. Les élus locaux dans la construction, l'explication. Et la construction de de de de de ces projets. Voilà je pense que la, la, l'efficacité, la performance de gestion des dossiers, elle est là et pas ailleurs. Que.

Il nous a trouvé tellement dans la Ligue mondiale qui va certainement investir en Espagne ou ailleurs. Donc la question. N'est pas de dire on va décider et le seul problème c'est la question administrative ou les délais administratifs ou les règles environnementales. La question est de créer un écosystème. Moi je partage ce que dit Franck besoin d'un récit mais de savoir là où on va. Qu'est ce que nous voulons produire. Quelle consommation sur quoi nous voulons re-acquérir une pleine souveraineté française ou européenne. Où j'ai envie de dire française et européenne. Comment recréer de la chaîne de valeur. Quelle formation pour les travailleurs et les travailleuses. Ce que disait Céline. C'est que c'est pas contre les collectivités. C'est avec parce que lorsque une entreprise veut s'implanter. Regarde d'abord si. Du coup, il y a un bassin d'emploi, est-ce que il y a des lycées professionnels et cetera où elle va pouvoir aller chercher des travailleurs et travailleuses quel service public. Elle va pouvoir offrir ses salariés, est-ce que ils sont Roms bien desservi en transports, vous voyez, c'est tout un écosystème. Donc la question et c'est pour ça que on vous l'a redit un certain nombre de reprises, à chaque fois on découpe, sujet par sujet, Alors qu'on a besoin d'avoir un débat global et donc la question de la réindustrialisation comme tant d'autres choses. Elle a besoin d'une réponse globale et de l'association. En priorité, des élus locaux et de la population et on ne peut pas se passer des deux, y compris de vouloir réduire les délais administratifs ou les enquêtes publiques c'est une bêtise. On a besoin de tout ça En ce sens qu'avec ce cet amendement, nous vous aurez interpellant et nous vous appelons à un grand débat public sur cette question. Monsieur le Sénateur, je ne retire aucun mot. Est ce que vous venez de dire. Et c'est exactement l'objectif de ce projet de loi. on travaille autant il y a des choses sur lequel le gouvernement et une immense majorité des sénateurs ne sont pas d'accord. Depuis un an, j'ai eu l'occasion de voir quelques discussions intéressantes sur le bouclier tarifaire, la finance des collectivités territoriales et cetera et cetera mais là-dessus, on est tous d'accord. On est tous d'accord évidemment que c'est un projet global et d'ailleurs dans le cadre de ses projets d'intérêts nationaux dans le cadre des débats publics dont nous allongeons la durée Monsieur le Sénateur gay on est réduit pas on les augmente dans le cadre de notre capacité à vouloir débattre de manière globale de zone industrielle globale et cohérente. Plutôt que de le faire briques de Lego par brique de Lego, tout ça c'est ce projet de loi qui permet de le faire et cet article, je le répète, il ne souhaite en aucun cas fragilisé la vie des collectivités territoriales et évidemment qu'seront associés comme c'est déjà le cas à l'ensemble des étapes de ces projets d'intérêt national. On souhaite juste. Pouvoir donner de la visibilité sur la procédure et on préfère que les collectivités territoriales qui s'opposera un projet le plutôt au début avant qu'on se lance dans un grand travail. Qui franchement mobilisera beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens au risque in fine et qu'il soit refusé. Faites-le au début. Plutôt qu'à la fin c'est tout. Merci monsieur le président. Bien. Je vais procéder au scrutin public sur ces trois amendements identiques de suppression. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du gouvernement les défavorable. Le scrutin public est ouvert.

contre 238. Ces amendements ne sont pas adoptés et je passe à 5 amendements en discussion commune le 175 monsieur bonhomme. Monsieur Bonhomme. Le 175. Merci Monsieur le Président. Oui je je présenterai amendement de mon collègue Pierre-Antoine Levi, qui propose donc de reconnaître la la raison impérative d'intérêt public majeur au projet concourant à la réindustrialisation. Et ce, au même titre que les projets d'énergies renouvelables pour qui cette reconnaissance a été consacré par la loi. À l'échelle de l'Union européenne, la Commission européenne a adopté un règlement temporaire en le 22 décembre 2022, dans lequel cette. Être affirmé À sécuriser juridiquement les projets en cas de contentieux lié à la demande de dérogation à l'obligation de protection stricts et des espaces protégés qui sont vous le savez, de retard et de difficultés. Cette mesure de simplification ne reviennent toutefois pas sur les conditions à remplir, en matière d'impact environnemental qui reste cumulative est obligatoire pour toute demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées. Merci.

au projet qui répondent à la double condition de souveraineté nationale et de transition écologique. C'est un argument qui qui s'inscrit dans le le débat que Fabien Gay appelle comme nous de ses voeux. Pour définir ce qu'est l'intérêt national majeur. Et et au passage je redis que la question de fond, le débat majeur, le débat des débats c'est celui de l'économie dont nous avons besoin pour réussir. Toutes les transitions nécessaires. Indispensables au monde vivable de demain.

et il vise à intégrer la dimension logistique dans les projets industriels pouvant être reconnue d'intérêt national majeur la réindustrialisation implique en effet le développement de sites logistiques qui accompagnent la production et le transport des biens ainsi manufacturés. C'est donc en toute logique qu'il faut les intégrer et intégrer cette dimension dans la qualification des projets industriels visés par les 2 alinéa de l'article 9. Merci le 299 Monsieur Merci monsieur le président, mes chers collègues. Cet amendement propose de supprimer le dispositif de qualification de projets d'intérêt national majeur à l'initiative des régions qui a été introduit en commission, nous comprenons bien une idée de marqué dans le texte la place prépondérante des collectivités locales dans la réindustrialisation. Nous souscrivons à cet objectif, qui est en réalité un état de fait que nous constatons sur le terrain. pose un double problème, d'abord d'un point de vue opérationnel ce dispositif mobilisera des ressources et du temps alors que l'esprit de l'article et du texte en entier et bien d'alléger les procédures et d'être plus compétitifs sur les délais d'implantation. Ensuite, et là c'est un problème institutionnel fondamental. Ce dispositif permet aux régions déterminer l'intérêt de la nation. Pourtant la Constitution dispose dans son article 20 que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Elle précise également son article 72 que que dans les territoires. C'est le représentant de l'État qui a la charge des intérêts nationaux. C'est pourquoi bien qu'en comprenant l'initier l'esprit d'encouragement à l'initiative que porte ce dispositif il nous apparaît pas opportun de le conserver. Hé bien de réaffirmer que l'intérêt de la nation est une prérogative du Parlement et de l'État.

à l'obligation de protection stricte des espèces protégées qui sont source de retard et de difficultés. Cette mesure de simplification. C'est important ne revient pas sur les conditions à remplir, en matière d'impact environnemental qui reste du cumulative est obligatoire pour toute demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées. Merci monsieur le rapporteur. Sur ces cinq amendements. projets d'infrastructures, le 147 sur les conditions cumulatives souveraineté et transition écologique le 359 sur l'intégration des chaînes d'approvisionnement. Le 299 sur la suppression de la qualification de projets d'intérêt national majeur par les régions. Pour vous dire que la procédure de mise en compatibilité créé par l'article 9 les très dérogatoire par rapport à la répartition normale des compétences entre l'État et les collectivités territoriales nous l'acceptons parce que certains nombres de cas qui devraient être extrêmement limités. Il ne semble pas opportun de l'étendre à davantage d'infrastructures aussi favorable soit telle et tout ça sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Je voudrais rappeler aussi à Monsieur Buy que ce n'est pas le président de région qui décident de de de définir une raison impérative. D'intérêt national majeur, ça reste le préfet en région qui pourra retenir sur la liste. Ces projets et les soumettre à cette définition. Ce n'est absolument pas le projet donc pour le le 175 sur les infrastructures, c'est une demande de retrait, mon cher collègue ou un avis défavorable pour le le par le le 175 pardon le 173 un avis défavorable pour le 147 c'était sur les conditions cumulatives on considère que ça réduit quand même considérablement le Champ des projets éligibles puisque s'. Des conditions. C'est donc un avis défavorable pour le 359 donc ça ouvre effectivement aux chaînes d'approvisionnement et la logistique. C'est donc un avis défavorable. Monsieur le Ministre, sur ces cinq amendements. et risquer du coup. Ben de passer de un 2 ou 3 projets dont je parlais tout à l'heure où à, à un peu trop ou pour le. 147 de réduire trop en introduisant une double conditionnalité là où nous souhaitions que ce soit, soit des enjeux de transition écologique soit des enjeux de souveraineté qui permettent de le faire donc défavorable sur tous ces amendements, sauf pardon, du sénateur Buy pour lequel le gouvernement est favorable. L'amendement introduit par la commission selon nous rallonge les procédures. Introduit un peu d'ambiguïté, je dirais, entre le rôle respectif de la région et de l'État et donc nous souhaitons revenir à la. Rédaction initiale, ce que propose l'amendement du sénateur Buy donc défavorable sur tout sauf le 299. Très bien. 175 2. Avis défavorable qui est pour.

Merci, monsieur le Président, je vous assure que j'avais la main levée mais je comprends que la présidence est un art difficile je je voulais faire une intervention parce que 2 de ses amendements proposent. supprimer la protection stricte des espèces protégées. J'ai été maire, j'ai eu des, ah que j'ai conduit aussi des projets d'aménagement et je sais très bien à quel point parfois la découverte d'une espèce protégée, nous fait craint de regarde des projets que nous défendons. Mais j'ai aussi travaillé avec des scientifiques de l'IP BES qui nous monte qu'à peu près un million de nos espèces sont menacées et que la disparition de ces espèces protégées dont on se dit parfois franchement ça n'est pas si grave peut avoir des conséquences qui sont des conséquences majeures. Donc je voudrais dire, il y a une tradition de dire on ne touche à la constitution que d'un doigt tremblant, je voudrais dire à tous les collègues on ne touche à la biodiversité que d'un doigt tremblant et plutôt on évite d'y toucher.

Rejeté le 147 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Rejeté. Le 359 de oui. Il a retiré il les retient. Le 299 avis défavorable de la commission favorable du gouvernement. Qui est pour.

Madame Billon. C'est un amendement de précision rédactionnelle qui vise à mettre en cohérence ses projets d'intérêt national majeur avec les objectifs de souveraineté nationale et de transition écologique qui vise à atteindre anticiper sécurisé faciliter tout projet d'implantation de nouveau site de production ou d'amélioration de performances industrielles, c'est l'objet l'industrie du futur, c'est aussi la production et transformation de matériaux matériaux stratégiques et bio-sourcés et bien entendu tout ceci n'est possible qu'avec la participation des collectivités. Je rejoins les différentes interventions de tout à l'heure et notamment de notre collègue Fabien Gay, ça ne pourra se faire cette anticipation cette sécurisation et cette facilité facilitation des projets que grâce aux collectivités, si elles sont intégrées à toutes les étapes des projets de leur conception à leur réalisation. Je vous remercie. Vous mentionnez là de de vouloir ajouter les secteurs stratégiques. Elle semble redondante. Par ailleurs il semblerait exagéré de considérer que tout projet améliorant structurellement la résilience économique de la France, peut être considéré comme concourant à la souveraineté nationale. Donc ce sera plutôt un avis défavorable. Si vous ne le retirez pas.

Que tout nous. Que comptez-vous faire sur la question de la formation sur le Ministre parce que j'entends, vous faites beaucoup de choses mais durant le premier quinquennat par exemple on a fermé les AFPA. Vous voyez. Et pour le coup, là ça permettait de former des milliers de personnes qui devenaient des salariés extrêmement bien formés et les pas pour l'instant elles ont pas été remplacés par grandes choses. 2ème question avec la réforme du lycée professionnel envisagé. Je vois une montée. Bouclier pas que du groupe communiste. Je vous rassure, d'abord des enseignants et enseignantes. Le lycée professionnel extrêmement inquiets mais aussi. Des élèves. Et les régions évidemment. Donc là il y a une question et puis la 3ème chose. OK pour réindustrialiser, bien évidemment, mais pas avec des emplois précarisés. Nous, nous voulons que ça accompagne. Avec des employes bien formés et donc bien reconnu et donc. Bien rémunérés et il y a une il y a une question autour de ça parce que la réindustrialisation et peut se faire avec un minimum de CDI et un recours massif à l'intérim ou au CDD. Vous voyez pas tout à fait la même chose et la dernière. C'est la question de la sous-traitance. Là il y a une question, il nous faut légiférer, je vous le redis, Monsieur le ministre, on a déposé une proposition de loi en ce sens. On l'a dit, on est prêt à travailler avec vous pour l'instant vous répondez pas mais sur la question de la sous-traitance en cascade. Il y a une vraie question et d'ailleurs on le voit sur les grands chantiers notamment sur les chantiers des Jeux olympiques. Je vous remercie. Oui, monsieur le président. Chers collègues, le la procédure créée par l'article 9 vise effectivement accélérer les implantations des traits des des très gros projet industriel et dans son premier alinéa ou le deuxième, ceux-ci sont déjà déterminées en raison, notamment, soit de l'importance de l'investissement soit en allant dans l'importance de l'emploi. C'est donc la question de l'adaptation des compétences en vue de la montée en gamme effectivement regrette que ce ne soit au travers la formation dans ce texte, mais pour autant nous le déplorons comme vous mais néanmoins considérant que c'est bien inscrit dans le, dans dans le dans les intitulés de l'alinéa de l'article 9 ce sera un avis défavorable. oui du gouvernement. Même avis très rapidement. J'entends ce que vous dites monsieur le sénateur, et une fois de plus, je suis d'accord avec presque tout ce que vous venez de dire. On a quasiment un million d'apprentis en France aujourd'hui, dont plus de 15% dans l'industrie, c'est un vrai succès de la formation à la française qui a transformé, non seulement le nombre mais surtout la qualité la mentalité. L'état d'esprit des Françaises et Français vis à vis de, de l'industrie, vous le savez, vous l'avez dit d'ailleurs les emplois industriels ça paye 22% de plus que dans les autres, il faut développer l'industrie, ce sont des emplois de qualité. Ce sont des CDI pour beaucoup. Les enjeux de la sous-traitance, je m'étais engagé à les échanger avec vous, il faut qu'on vous voit Monsieur le Sénateur dessus et donc je m'engage à vous recevoir pour évoquer tout ça mais là vraiment je pense qu'on est, je dirais, en dehors du Champ du projet de loi, même si on est sur un facteur extrêmement important, donc comme le rapporteur, un avis défavorable. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, avec tout le respect que je vous dois, on doit pas visiter les mêmes entreprises. Parce que là où m'expliquer où. Tout va bien dans l'industrie et peu de recours à l'intérim, aux CDD. Il y a qu'à aller voir dans les grandes boîtes. Non non mais dans l'automobile étant dans dans d'autres choses. Chaque fois que vous discutez. Avec des salariés mais aussi des directions le recours est massif. Le recours est massif à l'intérim et aux CDD. Non mais on a une vraie question parce qu'il y aura pas de réindustrialisation de ce pays sans des salariés bien rémunérés. C'est ça la une des clés c'est ça parce qu'une entreprise. C'est évidemment un patron des actionnaires. Nous vous savez ce que nous en pensons des savoir-faire des compétences. Et les travailleurs et des travailleuses d'ailleurs lorsqu'ils se mettent en grève. Il y a plus rien qui sort, donc c'est en 1er lieu les hommes et les femmes qui font vivre l'entreprise. Et donc là il y a une question. C'est que on ne peut pas avoir un projet de loi qui met au coeur la réindustrialisation du pays, sans parler du droit des travailleurs et des travailleuses. De leur compétence de leur qualification de leur rémunération. Vous me dites l'apprentissage est une grande réussite. C'est vrai que pendant très longtemps la dévaloriser. Non mais c'est une question mais les AFPA. Par quoi vous les avez remplacé la question du lycée professionnel, vous voyez bien qu'il y a un débat quand même et il faut réponde sur ces questions. Non mais je, je vous le dis ça et la question centrale aussi, vous voulez. Pas l'entendre. C'est la question de la sous-traitance. On a des grands chantiers. Non mais je reviens en ce moment les Jeux olympiques et le Grand Paris Express. C'est des grands chantiers pas industrielle au sens courant longtemps mais des grands chantiers. Là tu en es. Quel scandale. Quel scandale. Comme on exploite des gens y compris des travailleurs et des travailleuses sans papiers. Et des gens qui s'en lave les mains. Donc vous voyez ces questions elles sont intimement liés à la réindustrialisation notre pays. Donc si vous voulez pas longtemps on continuera à vous le faire savoir.

En parallèle avec le secteur du numérique. Aujourd'hui on peut se féliciter d'avoir une couverture. Par par la fibre. D'un d'un très bon niveau, mais à quel prix. Quand on regarde. À la fois je dirais les compétences de ceux qui interviennent les difficultés que l'on a aujourd'hui sur la la maintenant. Ces incidents à répétition. Le la la la faible le faible niveau de qualification de de la plupart des des des intervenants et des sous-traitants de niveau 1 de niveau de voire même de niveau 3 parfois. On a un vrai problème de compétence, on a un vrai problème de sous-traitance donc je crois que il ne faudrait pas que l'on répète ce ce ce schéma-là dans la réindustralisation. Parce que c'est tout aussi important, aujourd'hui, il est tout aussi important je dirais de de réussir la connexion d'une fibre que des pièces de très haute technologie ou. Dans, dans bien des domaines, donc. C'est un sujet c'est un sujet majeur le sujet de la formation. Le sujet de la sous-traitance qu'on ne peut pas négliger et qui doit aller de Pair avec tous les partenaires, que ce soit la région que ce soit les lycées professionnels, la formation, la formation continue. Tous ces points là ne doivent pas être étranger au au 10 discussions que nous avons. Qui est contre. Acheter. Le 353 Madame Paoli-Gagin. Merci Monsieur le Président c'est un amendement qui vise à intégrer des ouvrages de raccordement au réseau électrique gazier hydrogène dans le décret déterminant le périmètre des projets industriels intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition énergétique. Cette reconnaissance permettrait que les autorisations relatives au raccordement à ces réseaux d'énergie puisse être instruite dans les mêmes conditions de délais. Que celles relatives au projet industriel afin de ne pas risquer. De retarder en fait les 10 projets. C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir que le le décret couvrira bien les raccordements au réseau d'énergie. Nous avons besoin d'une garantie absolue sur ce point. Merci avait la commission. Oui, monsieur le président. Chers collègues, la commission a supprimé effectivement cette disposition figurant dans le texte initial qui permettait de faire bénéficier les réseaux de raccordement des projets d'intérêt national majeur des dérogations prévues à l'article 27 de la loi de l'accélération, c'est la dernière j'ai renouvelable une loi que nous avons voté il y a seulement quelques semaines. Elle comportait déjà d'ailleurs ce dans ce même article, des, des dispositions sur les leur car demain pour la décarbonation de l'industrie. Le gouvernement nous demande aujourd'hui de rouvrir le dossier. On aura l'occasion d'en reparler mais votre amendement ne permettra pas de toute façon de traiter les spécificités en matière d'autorisations d'urbanisme pour les réseaux électriques puisque l'article 9 vise à accélérer la mise en compatibilité des documents et non pas la délivrance d'autorisations d'urbanisme sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable. le gouvernement et et d'accord avec l'amélioration de la commission et dont souhaite plutôt le retrait de cet amendement et la préservation de la rédaction. Issue de la commission. Merci. Il est maintenu, madame Paoli-Gagin, il est. Il est. Ben justement le 363 à nouveau Madame Paoli-Gagin. Oui, monsieur le président. Les projets industriels d'intérêt national majeur devait également concerner la production ou la transformation de matériaux stratégiques et bio-sourcés, tant pour la résilience économique de notre pays que pour la transition écologique de nos sites industriels. Le bois, on l'a cité tout à l'heure et par exemple une matière première qui se décline en temps d'usage stratégique pour l'industrie, la construction, la distribution ou la production d'énergie. Cet amendement. Que je vous propose et de précision rédactionnelle et il vise à mettre en en cohérence ses projets d'intérêt national majeur avec les objectifs de souveraineté nationale et de transition écologique qui vise à atteint. merci monsieur le président. Chers collègues, la précision sans le sortir du Champ effectivement du décret du Conseil d'État visé par cet article qui a pour unique objet de définir succinctement succinctement ce que sont la transition écologique et la souveraineté pour préciser quel type de projets pourraient être qualifiées d'intérêt national majeur ce sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable.

Il nous faut mieux définir la notion d'intérêt général majeur et c'est donc le le propos de cet amendement 148 s'agissant ici d'une procédure d'accélération qui doit rester très exceptionnel. Nous proposons de conditionner la reconnaissance de la qualité de projets d'intérêt national majeur au projet de développement durable qui. Donc des garanties en termes d'empreinte environnementale de respect de la santé et de la biodiversité. Merci. Avis de la commission. Merci monsieur le président. Chers collègues comme vous l'indiquez, les profs, les projets d'intérêt national majeur resteront très exceptionnel. On a dit et le ministre-vient de le confirmer qu'il s'agirait d'un ou deux projets par an. Ces projets pourront concerner souhaite la transition écologique soit la souveraineté nationale ainsi qu'on dispose de texte de la la de lois la qualification de projets d'intérêt national majeur sera conditionnée. Je le redis, je viens de le dire à Fabien Gay. En terme de l'importance du projet en terme d'investissements, d'emploi et de superficie. Les critères que vous évoquez ont vocation à être évaluée dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet ainsi que le cas échéant dans le cadre de l'autorisation environnementale. Il ne me paraît pas opportun de les faire intervenir au moment de la qualification du projet comme projet d'intérêt national majeur puisque cette qualification n'emporte pas dispense des différentes procédures d'évaluation et de contrôle au titre du du code de l'environnement, ce sera donc un avis défavorable. il y a pas de régression dans cet article donc je suggère un retrait ou sinon un avis défavorable. Monsieur Montaugé. Oui je je j'entends les arguments qui viennent d'être développés. Bon on peut, J'en profite quand même pour. Réagir aux propos du rapporteur qui est et du ministre ailleurs qui qui nous disent et je comprends aussi que finalement il va y avoir peu de projets nationaux d'intérêt d'intérêt majeur. Oh ça je l'entends notamment par rapport au, au grand projet dont dont qui sont lancées, qui sont annoncés pour certains. Je voudrais, je voudrais profiter de de de de la parole pour pour attirer quand même votre attention sur la question de l'imbrication des chaînes de valeur. On peut avoir des petites entreprises. Dont on a besoin sur le territoire qui n'existent pas, qui veulent s'installer et caetera qui sommes partie prenante de la chaîne de valeur globale. De la, de, de la grande de qui a pu bénéficier de la notion de projet d'intérêt général majeur et et qui donc n'en bénéficieraient pas forcément moi moi je sais pas ce qu'il y a un sujet par rapport à ça, voilà ça, ça renvoie au au débat qu'on appelle de de de nos voeux par rapport à cette notion, moi je pense qu'on gagnerait

Très bien je mets aux voix cet amendement 148 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Acheter. Le 293 monsieur Merci monsieur le président je l'avais déjà évoquée dans ma prise de parole sur l'article. Cet amendement a pour objectif de prévoir le recueil de l'accord du maire et si nécessaire du président de EPCI préalablement à l'engagement de la procédure de mise en compatibilité instauré par cet article, nous considérons comme naturel que le maire ou le président de PCI dispose de leur pouvoir de décision s'agissant de l'accueil d'activité industrielle sur leur territoire. nous considérons qu'il faut recueillir cet accord au départ de la procédure, afin de les associer le plus étroitement possible en amont a fait parce que c'est eux qui connaissent le mieux le terrain et on ne veut pas perdre du temps inutilement par ailleurs conserver la demande d'accord en fin d'instruction instaurer un double verrou pouvoir avoir un effet des incitatifs pour les porteurs de projets. C'est pourquoi nous proposons de remonter le recueil de l'accord en amont de la procédure.

Peut être complètement différent de ce qu'il était initialement et pour lequel la collectivité a donné un accord si tout et qu'on construit avec les collectivités comme le gouvernement nous l'assure, il n'y aura donc aucune difficulté à obtenir in fine et l'accord des collectivités, un avis conforme concernés pour que soit adoptée la mise en compatibilité de leurs documents d'urbanisme. Je voudrais rappeler quand même ce que j'ai dit en propos liminaire, c'est que aujourd'hui on voit bien que l'organisation par exemple dans les Hauts-de-France. Qui n'est, qui ne devrait pas être de manière exceptionnelle a été une réussite. Aujourd'hui on voit que ce projet de loi, c'est d'essayer de prendre appui sur ce genre d'exemple pour coordonner accepté par toutes les parties prenantes. La réalisation de ces projets industriels majeurs. Moi je partageais complètement ce que disait madame brûle hein tout à l'heure, ce ne sont pas seulement les communes et les EPCI qui sont impactées certes pour les autorisations d'urbanisme mais pas pour la mise en conformité des documents d'urbanisme pour lesquels à la fois les départements au travers les infrastructures sont concernés et notre et en particulier la région quand même dans le cas de la modification du sera dette puisqu'elle a la stratégie en terme de développement industriel, il serait quand même assez étonnant qu'elle soit pas consultés pour accorder sa modification de son sera dette. Ça sera donc un avis défavorable. Vous l'avez bien compris. ensemble avec une procédure qui, je pense, permet de l'assurer, je profite de cette réponse pour répondre aux sénateurs Montaugé évidemment. Nous avons besoin des PME et des ETI pour fournir ces grands projets d'intérêt national. Mais si on n'a pas les projets d'national. Une chose est sûre, on n'aura pas les filières et on n'aura pas les PME, donc évidemment les PME les ETI vont bénéficier de l'ensemble de ces dispositions d'un texte, évidemment on doit s'assurer quand on crée une filière qu'elle fonctionne bien, il y a des filières en France qui fonctionne bien. L'aéronautique, on a des grands donneurs d'ordres qui sont prêts à à attirer et à prendre avec un certain nombre de PME de TI. Il faut que les nouvelles filières qu'on est en train d'installer en France photovoltaïque éolien. Le nucléaire évidemment que pas une nouvelle filière mais qu'on redynamise puisse tirer avec elle les PME les ETI, on s'en assurera mais cette. Procédure de projets d'intérêt national majeur, elle nous permet de créer des nouvelles filières en France. Allons-y, allons-y ensemble mais allons-y vite. Avis favorable. Mais on voit le 293 avec un avis défavorable.

Merci, monsieur le Président, votre Clément. J'ai entendu que Monsieur le Ministre s'arrête de de son propos. Simplement pour vous dire que cet cet amendement, nous sommes quand même empreint de bon sens car il paraît logique de recueillir l'avis de la du maire de la commune. Juridiquement compétente ou de l'EPCI juridiquement compétents suivant qui a la compétence urbanisme enfin ça nous semble être la base essentielle pour une acceptabilité du projet. Donc nous, nous pensons que cet amendement est plutôt empreint de bon sens.

j'ai j'ai des grandes ambitions pour Bernard. C'est pour ça. Là l'amendement de notre collègue Bernard buis enlève la vie de la collectivité tout au cours du processus que nous voulons, est ce que nous avons mis en commission et, pour le mettre que tout au début de. De du processus. Alors ce que dit notre rapporteur c'est que dans le processus de révision des documents d'urbanisme et dans le processus d'installation d'un projet, il y a plein de de modifications, il y a plein d'évolution des projets et nous, nous voulons que la vie des collectivités ils soient recueillies. Tout le temps en permanence c'est pas juste au début du projet. Voilà donc, attention à l'interprétation de cet admirable amendement mais pour lequel la commission est vraiment défavorable. Monsieur le ministre. Rapidement, donc ce n'est pas un amendement du gouvernement mais bien un amendement. Du sénateur Buy dont je rappelle qu'il est soutenu par l'Association des maires de France. Qui. Élevé. À juste titre contre la rédaction initiale qui je pense à travailler avec les élus notamment sénateur pour proposer cette rédaction qui permet aujourd'hui d'aller vite d'aller loin de le faire ensemble et qui n'enlève en rien évidemment les consultations des collectivités territoriales. Tout au long du processus, donc cet amendement, il est extrêmement bien, j'ai, j'aurais aimé que le gouvernement le fasse mais bravo monsieur bip pour cet amendement parfaitement rédigés extrêmement efficace.

dire un peu de confusion. Monsieur le rapporteur. D'abord, puis madame Maud Gatel. Oui, monsieur le président, Monsieur le midi je aurais pas laisser croire que l'association des maires de France n'a donné qu'un avis favorable à l'amendement de proposé par Monsieur Buy et pas par le gouvernement mais qu'il a donné aussi un avis favorable au nôtre. On a un mail en ce sens on pourra vous le fournir éventuellement. Bien merci de rajouter à la classe. Du débat. Madame Gatel. Merci Merci monsieur le président. On a l'air d'être dans le en même temps et je ne prétendrai pas. Apporter la lumière. Moi je suis embarrassé. Par cette affaire parce que je souscris au fait que. Un industriel a besoin de savoir si ça va être possible ou pas. Ce qui n'empêche pas de devoir respecter des choses. Je souscris au fait qu'il faut que les élus soient associés très rapidement et qu'il puisse dire, c'est possible. Chez moi, ou ça l'est pas, même si j'ai des exemples chez moi des projets qui ont eu toutes les bénédictions. Laïque et républicaine se sont vus contester à la femme malgré l'avis positif des élus par des militantes con on c'est bien le le chemin de croix de de ses affaires. Et en même temps, Monsieur le Ministre, si je puis dire mon embarras vient du fait que est-ce que ça veut dire que dès lors que vous avez interrogé demain président de PC que vous avez expliqué, il a plus rien à dire, même si le projet évolue. Donc moi je je je souscris à cette idée. De devoir en amont se prononcer parce qu'on ne peut pas balader les gens mais je suis quand même attentif, excusez-moi, je fais du en même temps. Maladroitement, mais quand même je suis attentif à l'alerte qu'adresse notre. Notre rapporteur là en plus, le président va dire je suis centriste. Donc je sais pas trop ce que je veux monsieur le président. Mais je voudrais juste trouver la lumière. Monsieur le Président, pour moi vous avez toujours été quelqu'un qui savait parfaitement ce que vous vouliez. Très bien. Non mais c'est. Vous savez, c'est le moment Monsieur Montaugé. Oui merci. Merci me monsieur le le président je je ne suis mandaté par personne pour faire l'exégèse des positions de l'AMF sur cet article 9. Mais moi ce que je comprends. Par rapport à ce qui a été dit, notamment par le rapporteur, c'est que ce sont des propositions de repli. Je voudrais le rappeler quand même et que la position de la notamment de l'AMF. C'est une position de rejet et donc de suppression de l'article 9. Bon. Allez, maintenant que tout le monde est éclairée. Je vais mettre aux voix donc le 293, avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement. Qui est pour.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers chers collègues. Nous considérons que l'article 9 est de nature à remettre en cause l'économie générale des documents d'urbanisme et donc, en cohérence avec l'article 1er du projet de loi qui organise la planification industrielle dans les sera Nous proposons d'associer un. Un monde de la qualification par décret d'un projet. Industriel d'intérêt national majeur l'ensemble des collectivités concernées par l'implantation de ce projet. L'acceptation locale du déploiement d'implantation d'industries vertes est essentielle à leur succès et aucune dérogation aux projets de territoire ne doit être autorisé ça l'accord des collectivités concernées. Donc il faut organiser la consultation avant toute prise de décision par l'État. Avis de la commission. Monsieur le rapporteur. une consultation de ces mêmes collectivités en vue de la qualification du projet. Comme intérêt comme projet d'intérêt national majeur cela alourdirait sans nul doute la procédure il sont plus pertinent que les collectivités soient consultés sur ce qui relève de leur compétence, à savoir la planification pour les régions et l'urbanisme pour les communes et les intercommunalités, ce sera donc un avis défavorable. Ah oui du gouvernement. Monsieur manteaux. merci Monsieur le le le président. J'entends les les les propos les arguments du du rapporteur. Je je peux les partager un un parti. Cela dit. La notion d'intérêt général majeur. Elle concerne absolument tous les Français. Voilà toutes les collectivités, et j'ai j'ai je ne vois pas pourquoi une une commune ne PCI. Départements et a fortiori une région ne serait pas associé. à la définition ou la qualification. De projets d'intérêt national majeur. Mais on voit le 150 avec 2 avis défavorable qui est pour.

En ceci qu'il intègre la possibilité de consultation des élus locaux pour leur permettre éventuellement de s'opposer à l'évolution de leurs documents de planifications cette évolution est très positif et conforme aux engagements que le ministre avait pris donc Monsieur le Ministre, le Sénat n'est pas ingrat. Je vous remercie de cette écoute et je remercie aussi la capacité de persuasion du rapporteur. Toutefois, on prévoit que les élus locaux puissent émettre des observations en amont de la procédure dans un délai d'un mois. L'autorité de l'État disposera elle d'un délai de 15 jours pour répondre, mais on sait que l'État ne reçoit pas toujours les courriers qu'on lui adresse et que ça veut dire que au-delà d'un mois, il est dit que la procédure pourra s'engager, même en l'absence de réponse de sa part. Vous comprenez que ça, ça n'est pas acceptable. Il y a un caractère absolument dérogatoire à cette procédure par rapport à la compétence aménagement donc nous nous demandons que l'État assure hein contradictoire et répondent de manière expresse aux autorités compétentes. C'est un préalable indispensable à la paisibilité de la concertation avec le public et Monsieur le Ministre, pour vous rassurer l'amendement proposé n'allonge pas les délais de procédure envisagée.

Défendu. Merci. Avis de la commission sur ces trois amendements identiques. Merci monsieur le président. Chers collègues, dans la mesure où votre votre pour vos propositions n'allonge pas les délais puisque le processus de mise en compatibilité peut commencer en parallèle. Dès que les collectivités ont fourni des observations, ce sera donc un avis favorable. Monsieur le Ministre, oui je je suggérerais plus. Tout un retrait, c'est bien la première fois que le Sénat. Nous propose à l'État d'être moins efficaces que ce que l'État propose lui-même nous on s'engage à le faire en 15 jours, vous nous donnez, à moi. Donnez-nous qu'un jour on y arrivera mais bon voilà plutôt retrait ou défavorables. Très bien je mets aux voix ces trois oui madame la présidente Gatel. Je voudrais pas être insistante et dire que je doute de la parole de l'État. Mais moi je pense que ce qui est dit doit être fait il est quand même dit que s'il a pas de réponse dans un délai d'un mois, les choses s'enclenche et que vous savez très bien monsieur le Ministre, ce que c'est le maire qui aura à répondre aux questions, aux interrogations. De de ses concitoyens et qu'il est très important qu'il est vraiment un argumentaire merci. hein. Non mais elle a quoi ça sert, lundi. Merci monsieur le président. Il ne s'agit en effet, pas seulement d'une question de délai parce qu'on pourrait dire chipoter pour 15 jours ça n'a pas beaucoup de sens au regard. De ses projets industriels qu'on, qu'on soit tous travailler mais l'idée c'est. Que l'État effectivement répondre aux observations remarque voire au au désaccord des élus sur un certain nombre de questions, vous nous permettrez. On est content que vous améliorer considérablement l'efficacité de vos services. Monsieur le Ministre, mais par expérience, nous n'avons pas toujours les réponses dans les délais où nous les attendons. Mais au-delà de ça encore, c'est ce qu'on a évoqué les uns et les autres tout à l'heure, c'est la nécessité d'un dialogue. Et d'éventuelles modifications des projets. puisse ils puissent. S'insérer convenir à tout le monde et c'est plutôt dans cet esprit-là que nous présentons ces amendements et d'ailleurs. Ne notre volonté de les maintenir et renforcer par l'amendement. Non pas du gouvernement mais notre collègue buis qui voulait en quelque sorte revenir sur. L'avis conforme des collectivités, ce qui est un peu contradictoire avec tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure Monsieur le Ministre sur votre volonté de vouloir associer pleinement les collectivités merci. je mais on voit ces trois amendements identiques, avec un avis. Défavorable du gouvernement est favorable bien entendu de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Ils sont adoptés. 2 amendements en discussion commune le 317 du gouvernement, monsieur le ministre. quartier. Monsieur le président. La la commission. A souhaité. Introduire une présomption. De qualification de raison impérative d'intérêt public majeur R IPM à tous les projets qualifiés d'intérêt national majeur sur le principe évidemment, nous considérons qu'il est très probable qu'un projet d'intérêt national majeur puisse profiter de ces qualifications. Mais je nous pensons que présumé par défaut cette qualification risque de poser un problème notamment sur l'équilibre environnemental de certains projets, la protection des espèces protégées et donc on considère pas qu'on doit en faire une règle générale comme la commission d'essayer de le faire et donc nous suggérons de restaurer une disposition qui me semble plus conforme à la Constitution qui était la rédaction initiale.

défendu. Ben voilà. Madame la présidente. C'est là où un long moment allez. Et j'en ai un troisième d'ailleurs en discussion commune. Monsieur le rapporteur. La 408. Oui, monsieur le président. En commission, nous avons introduit effectivement une présomption de reconnaissance de R de zipper M pour les projets d'intérêt national majeur dès lors qu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le gouvernement a bien voulu appeler notre attention sur le fait qu'il convenait que la loi encadre davantage la latitude laissée aux aux pouvoirs réglementaires de pour déterminer encore par en Conseil d'État par décret les conditions dans lesquelles un projet d'intérêt national majeur est réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur R 2 IPM. Afin de répondre à cet impératif constitutionnel. L'amendement précise la nature des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État pour permettre à certains projets d'intérêt national majeur de bénéficier d'une présomption de R 2, IBM, il s'agira de conditions. Dont rappelé l'importance monsieur Gay, c'est-à-dire les investissements et particulièrement l'emploi. Ces 2 paramètres sont déjà pris en compte pour qualifier un projet industriel d'intérêt national majeur cette disposition ne modifie pas par ailleurs la possibilité ouverte par le texte gouvernemental de reconnaître le caractère R 2 IPM à un projet d'intérêt national majeur dans le décret qui le qualifie comme telle en fonction des caractéristiques propres y compris, si les conditions fixées pour bénéficier de la présomption d'de R 2 IPM ne sont pas satisfaits. Monsieur le rapporteur. Tant que vous y êtes, donnez-nous l'avis de la commission sur l'amendement du gouvernement et sur le 287. Alors je vais me répéter un petit peu nous avons introduit donc cette présomption de reconnaissance 2 IPM pour les projets d'intérêt national majeur dès lors qu'ils se satisfont à ces conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cela nous semble justifiée, étant donné l'ampleur des projets. Ils sont d'ailleurs jugés suffisamment important pour justifier des dérogations exorbitante à la répartition des compétences entre collectivités. Vous aviez d'ailleurs me semble-t-il. Monsieur le Ministre souhaiter que l'ensemble des projets d'intérêt national majeur bénéficient d'une présomption de R 2 IPM. C'est en tout cas ce qui figurait dans l'avant-, projet de loi à nos collègues écologistes je signale que rien ni dans le droit européen ni dans la charte de l'environnement ne faisait obstacle à ce que la loi définit des critères permettant de considérer que certains projets répondent à une raison impérative d'intérêt public majeur. Le Conseil d'État a eu l'occasion de le préciser, notamment à l'examen du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Je rappelle également que le R 2 IPM n'est que l'une des conditions pour accorder une dérogation espèces protégées. En ce qui concerne les 2 autres amendements j'ai expliqué, la manière dont notre amendement prend en compte la remarque du gouvernement. Ainsi le pouvoir réglementaire hé bien encadré cet encadrement reste cohérent avec la nature des projets d'intérêt national majeur je précise donc à nouvelle à nouveau pardon que cet encadrement ne fait absolument pas obstacle à l'autre mesure sur la R 2 IPM prévue à cet article par le gouvernement, à savoir la possibilité pour le Premier ministre après un examen au cas par cas de reconnaître à un projet d'intérêt national majeur dans le décret qui le qualifie comme telle afin de purger le contentieux sur ce point. Au début des projets. Ce sera donc Monsieur le Président, un avis favorable pour l'amendement 408 est défavorable pour l'amendement 317. enfin, de 400, c'est le vôtre. Heureusement que c'est favorable mais. Le trois 17 et le 287 les sur les deux, vous êtes défavorable. Donc Monsieur le Ministre. Alors si vous me dites que vous êtes favorable aux. J'allais dire mais finalement je vais m'en passer la demande je vous dire que j'ai été presque favorable à l'amendement de me. Ce excellemment défendu par ailleurs en fait il est très proche d'une autre. Mais le nôtre et et je dirais permet d'avoir une coordination avec la ligne à 23 donc je préférerais le notre vote mais si vous voulez voter le nôtre, n'hésitez pas et de ce fait. Défavorable aux 408 qui résout une partie du problème mais pas l'ensemble, vous l'avez dit, nous l'avions dans notre avant-, projet de loi proposé cette disposition, le Conseil d'État nous alerter sur le fait que c'était sans doute un anti-constitutionnelle. Vous l'avez rétabli vous l'a précisé dans l'amendement 408 mais je, j'ai bien peur que ça ne suffisent pas et que ça laisse toujours. Une disposition anti-constitutionnelle donc opposé au 408 est favorable, évidemment celui du gouvernement est défavorable ou retrait à celui de monsieur Très bien. Alors je mais aux voix à Monsieur Gay. Hé oui on a fallu. Monsieur le président je je retire le nôtre au profit de celui du gouvernement. j'espère que ça va être noté dans le procès-verbal. Si. Mais vous faites une promesse. Vous regardez vous regardez pour augmenter les salaires des travailleurs. Non mais attendez, là on va en rester aux amendements hein allez donc d'abord le 317 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Merci. Et qui est contre. Il est adopté et il fait donc tomber le 408. Et je passe au 318 du gouvernement. Voilà. Le 318 du gouverneur dans. Il s'agit. Mais monsieur le président de rétablir des dispositions prévues par le projet initial supprimé en commission concernant le raccordement électrique des projets d'intérêt national. Objet de l'article 9, le raccordement électrique est évidemment un des éléments essentiels de ces projets. Les industriels nous le disent tous, ils veulent du foncier. Des calendriers et de l'électricité décarbonnée pas cher. Ça tombe bien, on en a en France, assurons-nous qu'ils l'ont en temps et en heure. Merci. comme tout à l'heure qu'. Une, je l'ai dit nous avons supprimé en commission les dispositions permettant au réseau de raccordement des projets d'intérêt national majeur de bénéficier des larges dérogations prévues à l'article 27 de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, que nous avons adopté il y a seulement quelques semaines, on revient dessus. Nous trouvons sur le fond vous souhaitez permettre à l'État de modifier l'ordre de classement des demandes de raccordement pour garantir un raccordement rapide des projets d'intérêt national majeur. On peut l'entendre, c'est l'article 28 de la loi ENR je note tout de même que cette sorte de classement ne peut être modifié que si le délais de raccordement de l'un des projets sur la zone donnée est supérieur à 5 ans, c'est un peu long pour les projets dont nous parlons, je ne suis pas convaincu de l'efficacité de la mesure en ce qui concerne l'article 27 de la loi et nerfs. Il prévoit de larges dérogations en matière de participation du public d'évaluation environnementale de protection des sites et paysages remarquables et des milieux à préserver de telles dérogations qui sont exorbitantes sont-elles vraiment justifiées pour les projets industriels d'intérêt national majeur, l'étude d'impact reste indigente en outre l'article 27 de la loi et nerfs dans sa rédaction actuelle permet la mise en oeuvre de ces dérogations pour une durée limitée, 2 ans renouvelable au maximum une fois mais dans la rédaction que vous proposez cette limite de temps ne s'applique pas au raccordement des projets d'intérêt national majeur, ce n'est donc pas un simple décalque des mesures prévues à l'article 27 de la loi sur les énergies renouvelables, cela va bien plus loin. On le voit bien, il n'est pas de bonne politique que de légiférer dans la précipitation vous rouvrez une loi votée il y a quelques semaines. Faites-nous des propositions équilibrées et on pourra sûrement en rediscuter. Ce sera donc un avis défavorable. Mais aux voix l'amendement 318 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Je mais aux voix l'article 9. Qui est pour.

Le 134 Monsieur Salmon. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. L'article 9 bis adopté en commission prévoit que l'artificialisation des sols liés aux installations industrielles ainsi qu'aux équipements et logements à soient exempts du décompte Dusan. Tout d'abord, nous ne pouvons souscrire à ce dispositif sur la forme car il anticipe sur les débats. Les travaux en cours à l'Assemblée nationale où la proposition de loi sur la mise en oeuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols n'a pas encore été voté, c'est ce véhicule législatif qui doit déterminer les modalités précises de comptabilisation notamment pour les projets d'envergure nationale. Sur le fond, notre groupe défend la mise en application des objectifs du zéro artificialisation nette et reste bien entendu cohérent sur sa ligne. Le rythme d'artificialisation de nos espaces naturels agricoles et forestiers est absolument insupportable. Ils remettent en cause notre autonomie alimentaire la biodiversité de nos territoires. Nos capacités de stockage de carbone une prise de conscience était déjà à l'oeuvre sur le caractère intenable en ce modèle de ce modèle de développement sur la nécessité de réduire la consommation des Hénaff. Sur la réindustrialisation. Si elle est nécessaire pour des questions de transition écologique et de souveraineté les projets industriels n'ont pas à être exonérée de cette trajectoire Dusan car il participe bien au recul des Terres agricoles et des espaces naturels dont nous avons besoin pour préserver la biodiversité. Il n'est pas question de mettre l'industrie en dehors de la société en dehors de la biosphère. Cela ne doit pas non plus directement l'enveloppe de la commune d'implantation, afin d'éviter la double peine pour les Thierry victoire qui seraient privés d'une très grande part de leur capacité à agir à cause du poids des infrastructures nationales. C'est pourquoi, ces projets doivent être recensés au sein d'une enveloppe nationale et le décompte des surfaces artificialisées doivent ensuite être répartis de façon équitable entre les régions. Je crois qu'il y a des débats ce sujet au niveau du gouvernement. Merci. Merci monsieur le président, chers collègues. On a mis en conformité, je dirais l'application de la loi than quoi. La PPL telle que nous l'avons voté ici dans cette loi industrie verte vous comprendrez donc que c'est un avis défavorable Il est favorable. Je reconnais que le gouvernement a eu quelques débats sur ce sujet extrêmement important mais le gouvernement désormais ne fait plus qu'un. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la discussion et la rédaction qui est issu de la commission à l'Assemblée nationale qui doit encore faire l'objet d'un vote en séance, je le reconnais bien évidemment d'une discussion en commission mixte paritaire puisse conduire les sénateurs à vouloir comme on vous disiez madame la présidente. Non non c'était une assurance vie aussi dont vous parliez l'autre fois, une assurance vie sur la PPL issu du Sénat mais mais telle qu'il est rédigé au aujourd'hui cet amendement je dirais nous fait revenir en arrière par rapport aux avancées de l'Assemblée. Nous considérons évidemment que le débat doit pouvoir se poursuivre à l'Assemblée, je l'espère obtenir une conclusion conclusive, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, dans le cas de la commission mixte paritaire, donc nous sommes favorables à cet amendement du sénateur seulement qui permet au débat de se poursuivre à l'Assemblée et une autre d'avancer. Merci. Madame la présidente. Oui, merci Monsieur le Président. Je veux d'abord dire à monsieur seulement qu'on n'est pas là dans le climat contre. L'industrie. On est là sur un projet d'industrie verte sur des panneaux photovoltaïques sur des éoliennes sur des batteries qui vont nourrir la transition écologique. sur des grandes infrastructures de transport qui vont aussi normalement nourrir la transition environnementale telle qu'on la souhaite tous donc on essaie de pas opposer les choses. Monsieur le. Monsieur Salmon. La la 2ème chose. Vous l'avez parfaitement analysé. Monsieur le Ministre. Pour l'instant, peut-être que le gouvernement a trouvé un accord entre les différents ministères. Mais pour l'instant c'est le Parlement qui est en train de discuter et donc tant que le Parlement s'est pas mis d'accord dans le cas d'une commission mixte paritaire et trouver un accord qui répond aux objectifs à la fois de cette loi mais aussi des différents objectifs qui ont été poursuivis dans la proposition de loi Hazan ici voté très largement, je le répète, au Sénat, hé bien nous n'avons pas de certitude donc comme la commission mixte paritaire sur l'industrie verte n'aura lieu qu'à l'Automne pour des raisons de calendrier législatif. Voilà ben bien sûr et puis comme ça on aura le temps de regarder le PLF, et de voir si vous êtes au bout de vos obligations hé bien. On verra dans cette discussion de CMP qui sera. CMP than. Si on a obtenu satisfaction. Voilà donc comme vous l'avez dit, je préfère prendre une assurance vie. À ce moment. Merci monsieur le président, mes chers collègues, Lausanne et bien évidemment une question centrale pour notre industrialisation puisque le foncier est une condition nécessaire à l'installation d'activités industrielles. Nous comprenons la position du rapporteur et de la présidente de la commission mais nous semblons privilégier un compromis qui pourrait être trouvée et aujourd'hui nous sommes favorables à cet amendement de suppression car oui un hectare artificialisés même pour de bonnes raisons doit compter, nous souhaitons que ce compromis soit confirmé en séance et adopté dans une future CMP, c'est pourquoi nous soutenons aujourd'hui la suppression de l'article 9 bis qui exclut l'industrie mais également les prix aménagement et qui peut m'a besoin en logements qu'elle suscite du décompte Dusan et nous semble aller trop loin et nous privilégions donc le compromis qui pourrait être. Abouti prochainement. Oui, monsieur le président. C'est juste pour rebondir sur les propos de madame la présidente de la commission des affaires économiques. Nous non plus nous ne sommes pas là pour opposer la réindustrialisation la relocalisation et l'environnement. Bien entendu, on a besoin de réindustrialiser. On pourrait revenir sur la définition de l'industrie verte, mais je ne vais pas le faire, ça prendrait encore un peu plus de temps simplement, est-ce que lorsque l'on implante une industrie on artificialiser. Oui donc il y a artificialisation donc ce doit être décompté quelque part au niveau national pour nous et après, avec une péréquation au niveau des différentes régions Dire que ben, parce que c'est de l'industrie ça n'. Lisent pas parce qu'on en gros si on regarde mot mot voilà ce que ça voudrait dire hé bien non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réalité. Donc regardons les choses en face et comptabilisons sept artificialisation de l'industrie. Merci. Merci je suis saisi d'une demande de scrutin public sur cet amendement par le groupe écologiste. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable que l'avis du gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56, le scrutin est ouvert.

Demande voter le scrutin est clos. En 343, exprimés, 263 pour 50 contre 213. L'amendement n'est pas adopté. Et je passe un amendement 319 du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci. L'objectif il est, pour les mêmes raisons d'ailleurs de supprimer l'article 9 bis et de renvoyer vers les débats en cours dans le cadre de la PPL sénatoriale. Madame la présidente évidemment loin de moi l'idée de De prendre la place du Parlement, Assemblée et Sénat réunis sur sur ces débats. Donc je comprends tout à fait la logique de vos amendements ces amendements de suppression nous permettent au gouvernement d'afficher.

Sous-amendement Madame Paoli-Gagin le 409. Merci monsieur le président. Ce sous-amendement vise à préciser l'amendement du gouvernement. Pour indiquer que la loi mentionné par le dispositif de l'amendement doit aussi exclure les ouvrages de raccordement au réseau des calculs, des surfaces artificialisées dans l'objectif Dusan. Les renforcements de réseaux sont nécessaires au raccordement industriel et à la sécurité d'approvisionnement énergétique. Merci. Avis de la commission sur l'amendement et le sous-amendement. Oui, merci Monsieur le Président. Alors votre amendement. Monsieur le ministre effectivement mieux disant que votre texte initial mais il est beaucoup moins disant ans que ce qu'il dit l'article 9 bis que nous avons rédigé introduit par notre commission, il oublie toutes les infrastructures, notamment celles qui viennent d'être précisés liés aux implantations industrielles, mais aussi les logements pour les salariés. Je donne donc un avis favorable au sous-amendement 409 qui va dans le sens de nos propositions. Il oublie aussi de les très grands sites que vous comptez près équipée. S'ils ne trouvent pas preneur l'artificialisation en sera-t-elle imputés aux collectivités d'implantation. C'est une question. Par ailleurs, la loi fait bien ce qu'elle veut et vous le savez donc bien que votre rédaction fait reposer l'exclusion du zen sur une hypothétique loi à venir. On vient d'en parler. La PP alezane. Si seulement elle aboutit, elle n'a donc aucune valeur juridique. Elle ne donne comme l'a dit la présidente Prima aucune garantie. C'est pour ça qu'on prend une assurance elle donne certes un bon signal en prévoyant explicitement l'exclusion Dusan de l'ensemble des industries de la chaîne de valeur des activités dans les secteurs du développement durable. Mais elle peut aussi d'un autre côté inquiétés en ne mentionnant que l'exclusion des objectifs chiffrés locaux et non régionaux et laisse donc la porte ouverte à la mutualisation dont nous ne voulons pas je Béchu nous promettait en mars que la question soit réglée dans le texte sur industrie verte. Monsieur le maire nous dit à présent qu'elle le sera dans la PPL than en bref trop d'incertitudes et un amendement qui ressemble à un marché de dupes. Ce sera donc un avis défavorable. Monsieur le Ministre, votre avis sur le sous-amendement. Donc je comprends que le Sénat veuille s'assurer que la main et garder sur les débats jusqu'à la commission mixte paritaire, je tiens à vous assurer en tous cas que le gouvernement soutient le processus de l'Assemblée telle qu'il est arrivé à ce stade, y compris un sous-amendement qui je pense va rassurer la sénatrice. Paoli-Gagin pardon. Donc voilà. Demande de retrait sur le sous-amendement. Bon on est bien d'accord. La commission est défavorable à l'ensemble. C'est un peu curieux parce que favorables sur le sous-amendement mais défavorable à l'amendement. Ça n'a pas beaucoup de sens. Pardon de vous le dire mais bon. Commençons par le vote sur le sous-amendement 409 avec, si je comprends bien un avis défavorable du gouvernement favorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Je crois que plus personne. Oui très bien. Il est. Adopté. Donc je passe à l'amendement du gouvernement. Ainsi sous-amendé. Avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Bon donc. Tout ça est rejeté. Merci beaucoup. 5 amendements en discussion commune le 200 très il y a 3 identique d'abord le 213. Madame Joseph. Oui, monsieur le Président, cet amendement de monsieur d'arrêt Sautarel. Disent ainsi exclure du décompte Dusan des collectivités d'implantation, y compris les régions, les projets de production d'énergie renouvelable en effet ces installations contribue à l'arrêt Alisa Alisa sur des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et concourent à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation, l'objectif de cet amendement est ainsi de ne pas contraindre les collectivités en charge de l'aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets, de production d'énergies renouvelables et des projets d'aménagement de locaux. Merci. Le 335 madame Paoli-Gagin. Il est défendu monsieur Prix. Merci. Le 386 n'est pas défendu 14 à nouveau deux amendements identiques à nouveau Madame Joseph. Sur le 214. Oui donc cet amendement de monsieur tout à fait légalement vise c'est un amendement de repli. Qui vise à exclure du décompte Dusan des collectivités d'implantation, y compris les régions, les projets de production d'énergie renouvelable relevant donc d'une ère IPM afin de ne pas contraindre les collectivités en charge de l'aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets, de production d'énergies renouvelables et des projets d'aménagements locaux parce que la reconnaissance de la. Pour ses projets de ENR leur confère une dimension d'intérêt public. Merci. Le 387 n'est pas défendu. Avis de la commission sur les trois amendements soutenus. excluez de les faire bénéficier d'une exemption than. Nous n'avons pas non plus jugé utile d'inclure dans notre PPL alezane ce cet élément votée en mars dernier par souci de cohérence dans ce qu'on a voté. Ici au Sénat, ce sera donc un avis défavorable pour les amendements de 113 335 286. Je l'ai oublié celui qui n'était pas défendu et le fait que les projets concernés soit reconnu avoir le caractère de projets répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur qui concerne la dérogation espèces protégées ne change rien à l'affaire. La vie et des également donc défavorable pour les amendements, 214 et 387. Du gouvernement. Très bien je mais aux voix les 213 et 335 identique avec 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Rejeté. Ensuite les 2 identique. Enfin, le seul qui reste le 214 avec à nouveau deux avis défavorable qui est pour. compte. Acheter. Le 354 madame Paoli-Gagin. Il s'agit d'un amendement qui vise à exclure les ouvrages de raccordement au réseau des calculs, des surfaces artificialisées dans le cas de l'objectif en cohérence avec les amendements précédemment déposée. Merci. Avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le Président. Votre amendement est satisfait par là l'idée à 9 de l'article 9 bis puisqu'il prévoit également une exemption Dusan pour les équipements liés au projet industriel exemptés Dusan ce sera donc une demande de retrait, le cas échéant d'avis défavorable.

Et l'article dans son intégralité puisqu'il concerne uniquement les projets mentionnés, l'article 9 de la présente loi, nous souhaitons nous étions donc distinguer ces projets à caractère industriel de l'ensemble des autres projets qui pourraient entrer dans une enveloppe nationale alors cette disposition. Elle est d'ailleurs déjà prévue par la petite IV de la PPL sénatoriale relative aux objectifs du zéro artificialisation nette adopté au Sénat, en mars dernier qui s'étendra au projet d'ampleur nationale, ce qui nous concerne pas uniquement les industries alors pourquoi faisons-nous cette proposition dans sa rédaction actuelle. L'article 9 bis ignorent les conséquences de l'artificialisation entre guillemets une bonne et une mauvaise a. Artificialisation une que nous pourrions laisser faire sans la comptabiliser qui concernerait les industries et une mauvaise qui concernerait nos collectivités déjà très pénalisés. Puisque ayant très peu artificialiser. Si ces 2 exemples ne peuvent évidemment pas être traités à l'identique et ce n'est pas ce que nous proposons. Il est en revanche urgent d'entendre l'impératif écologique et son actualité brûlante, la biodiversité, le dérèglement climatique ne regarde pas si l'imperméabilisation des sols et fait part des projets nationaux ou locaux. Et il est nécessaire de tendre vers un équilibre entre artificialisation et des artistes suffit. Signalisation avec la création d'une enveloppe nationale qui contribuera aussi à la prison, même par l'état des objectifs qu'il impose aux collectivités merci avait de la commission. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, chers collègues. Prévoir une comptabilisation séparé au niveau national revient à mutualiser l'artificialisation induite entre les régions. La mesure d'exemption perd ainsi tout son intérêt. C'est comme en double comptabilité financière hein. La double comptabilité foncière ne vaut rien puisqu'à la fin, rien ne se perd, rien ne se crée, c'est comme le débit et le crédit. Par ailleurs reconstituer le montant des surfaces artificialisées par des projets industriels, sur les 10 dernières années serait un travail de fourmi qui excède sûrement les capacités de l'État et des collectivités, l'État ne peut même pas nous fournir pour les seuls projets publics. Je vous propose d'en rester un dispositif simple et clair de nature à restaurer à rassurer pardon tant les porteurs de projets que les collectivités et je vous rappelle qu'on a proposé, on propose un rapport d'étape dans trois ans, qui nous montrera c'est certain que l'exemption Dusan pour les implantations une industrielle n'aura pas fait déraper la trajectoire nationale ce sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Même avis du Gouvernement je mais au voit le 251 avec 2 avis défavorables est pour.

Moi je ne crois pas que la stratégie industrielle, c'est seulement. L'attractivité des investissements étrangers ou on est très attractif, très bien, on s'en réjouit mais c'est un peu différent d'une politique de réindustrialisation, une souveraineté parce que lorsque il y a des investissements étrangers. Ça veut dire que la prise de décisions politiques et industriels. Elle se fait pas en France elle se fait à l'étranger. Et donc on n'est pas sur une compétence de souveraineté et pardonnez-moi de vous le dire. Pour l'instant le bilan aussi suivant. Souvent vous l'oubliez mais enfin la vente de fleurons industriels aux étrangers Nokia Technip. Je rappelle pas la branche. Électrique d'Alstom Hadji. Les chantiers de l'Atlantique et tant d'autres choses. C'est ça votre bilan quand même. La vente de fleurons industriels. À l'étranger. Donc il y a une question, oui à l'investissement étranger mais faut garder quand même. Une zone de contrôle notamment parce que pour attirer ses voeux investisseurs étrangers. On le rappelle pas assez souvent nous sommes champions du monde d'argent public pour accompagner le capital ben oui. Oui oui oui oui oui oui oui. 160 milliards d'euros chaque année. Ben oui mais il faut le dire. Non mais quand on a un débat politique. politique. Le ministre, il ne faut pas prendre un argument et oublier le reste, 160 milliards d'argent public dépensés chaque année pour accompagner le capital. C'est bien loin de ce que les travailleurs et travailleuses engrangeant salaire. Et bien loin aussi de ce qu'engrange des actionnaires beaucoup plus élevé. Donc nous, nous proposons une chose. D'accord pour accueillir des. Investisseurs étrangers mais on veut étendre la zone de contrôle et notamment on aura un débat ensuite dans l'autre partie sur le remboursement des aides publiques lorsqu'ils s'en vont donc en nous proposant. Au minimum, de renforcer le contrôle sur ces investissements étrangers je vous emmerde. Merci monsieur le président, chers collègues. Pour ce qui est de la souveraineté nationale votre amendement et heureusement satisfait par le droit existant. Pour ce qui est de la transition écologique. Il me semble que le pouvoir réglementaire ferait en effet bien de considérer certaines activités critiques comme relevant de la souveraineté nationale pour autant votre amendement semble assez problématique car d'une part comment vérifier quel projets auront bénéficié des dispositions de la loi sur l'industrie verte. Comment tenir compte. Raconte pardon des usines qui auront bénéficié de la part parfois de petites communes du déclaration de projet par exemple. Il ne s'agit pas de faire le suivi de subventions ou d'un crédit d'impôt, la mesure ne semble donc difficile à mettre en oeuvre. D'autre part nous cherchons pour l'heure à attirer des investisseurs étrangers qui ne vous effraie pas, d'ailleurs vous l'avez dit. Dans les secteurs de la transition écologique, c'est ce que vise en particulier l'article 9 ne risque-t-on pas justement de les effrayer. Avec une telle mesure. Je ne vais pas prendre l'exemple mais on pourrait citer les les les celles qui viennent de s'installer dans les Hauts-de-France. Bref je souscris à l'intention que vous que vous dites j'invite le gouvernement à y réfléchir mais votre dispositif me semble présenter un risque important d'effets de bord, ça sera donc un avis défavorable. Vous contredire vous avez une Coupe du monde de retard. Je veux dire l'inflation réduction Act des États-Unis, là on change de dimension. Les pourcentages d'aide dont on parle dans le cas de ce projet de loi les pourcentages d'être dans lequel dont dont on parle dans le cas du du programme. France 2030, c'est 25 à 30% d'aide sur des investissements sur seulement l'investissement en capital en machine des investisseurs qui viennent nous rejoindre. Aux États-Unis, on a changé dimensions il finance tous les machines et les opérations et cetera, moi je pense personnellement qu'ils vont très loin. Sans doute un peu trop loin. On est aujourd'hui cohérent et concurrents et compétitif en termes de Tolède, avec nos partenaires qui parfois son concurrent européen. Et on met en place un certain nombre de dispositions dans le cas de ce projet de loi pour nous remettre au niveau mais. On est peut-être sur le podium. On est loin d'être champion du monde. Sur le contrôle des investissements étrangers en France. Ce projet de loi et vise à accélérer les installations en France de nouvelles usines. Et ce à quoi vous faites référence c'est des installations des entreprises d'ores et déjà présente en France qui ferait l'objet de procédures d'acquisition par des investisseurs qui finalement plutôt que de venir construire des usines préférait les. Quelle voire même parfois avec un risque qu'les dès la colline elle elle relocalise chez eux donc le contrôle des investissements étrangers en France, c'est une préoccupation extrêmement importante de ce gouvernement et j'allais dire de la majorité actuelle à l'Assemblée et de la majorité précédente et je pense que là-dessus, on s'est retrouvé avec la majorité du Sénat la présidente Prima s'en souvient. Dans le cas de la loi pacte. On a élargi par le décret donc élargi le Champ du décret dit I E F investissements étrangers en France qui permet d'élargir notamment aux secteurs qui. Mettent en danger la souveraineté nationale, le contrôle du gouvernement et sa capacité à refuser des investissements donc non seulement votre amendement. Il est satisfait, je souhaite rappeler que le ministre-Bruno Lemaire a prolongé le taux de pourcentage de détention minimum qui fait que l'État a son mot à dire si un investisseur étranger et détient plus de 10% d'une entreprise ou souhaite pardon. Détenir 10% d'une entreprise ou plus. Donc nous considérons qu'elle est couverte par le décret AUF l'État peut mettre en place la procédure d'investissements étrangers en France et éventuellement s'il le juge utile soit mettent des conditions soit refusé l'opération donc je pense que cet amendement il est largement respecté donc je suggère un retrait.

Les Américains c'est produire américain. Et consommer américain et soutien à la production et à la consommation américaine. Et donc retour sur investissement, investissements dans le savoir-faire dans l'outil dans les compétences et y compris l'investissement productif sur le long terme, donc avec un retour. Pour le territoire national, nous c'est pas ce qu'on fait. Il y a aucune contrepartie de rien. 160 milliards mis sur la table. Et j'entends ce que me dit monsieur le rapporteur. Ça serait trop compliqué. On va. On ne va pas réussir à contrôler et cetera mais enfin bon quand il faut contrôler l'argent public. Par exemple pour le droit des allocataires chômage là il y a pas de problème, on est capable d'inventer, y compris bien savoir où c'est fléché. Et y compris le pouvoir sanctionner. Par contre, lorsqu'on parle de l'argent donné au capital dans ce pays. Alors là tout impossible. C'est infaisable. Et donc je vous le dis. Les 160 milliards donnés chaque année. On n'est pas sûr que ça aille dans l'investissement productif dans les compétences et dans les salaires. Par exemple le CICE. Non mais parce que quand même on a on a un retour d'expérience sur un certain nombre de choses. Le CICE et c'est pas le groupe communiste qui le dit c'est services du Premier ministre, c'est je ne sais plus combien. Près de 400.000 euros par emploi subventionné.

Merci monsieur Montaugé. Et. Merci Monsieur le Président. Les sujets de Downtown, débat à l'instant sont sont fondamentaux. les Américains. Ont pris des options stratégiques lourdes comme il l'avait fait d'ailleurs par le passé notamment pour accompagner. L'écosystème numérique avec le succès que l'on sait.

Vont être dans une situation. Comparable. À celle. Des entreprises qui vont être accompagné aux États-Unis dans le cadre de l'IRA. Voilà parce que c'est cette question là de de la réponse à cette question-là. Va dépendre. L'avenir économique, social et même environnementale. De notre pays et et du continent européen dans le cadre à la concurrence internationale. Des des de la globalisation. Mondiale. j'ai j'ai on a jamais eu l'occasion d'aborder ce ce sujet en tout cas comme ça aussi aussi directement mais je crois que c'est cette question là elle est absolument fondamentale pour l'avenir de notre pays et pour la souveraineté puisque c'est c'est quelque part l'objet l'objet de cet amendement de de notre de Monsieur le Ministre. Vous souhaitez. Crédit impôt-recherche. Nous considérons que c'est déjà conditionné par de l'innovation et de la recherche et là encore. Un élément important de la compétitivité du site France. Mais sur ce que vous mentionnez là sur France 2030. Tout ça est extrêmement conditionné tout ça est extrêmement rigoureusement analysé par les services de l'État par les services de la Commission européenne et les subventions industrie verte c'est pas des chèques en blanc c'est vraiment des chèques envers qui permettent d'accompagner des investissements de qualité conditionnée à la décarbonation soit de l'industrie traditionnelle, soit de la mise en oeuvre des nouvelles industries et donc de ce point de vue là je pense qu'on peut se retrouver concernant la la question du, du sénateur Montaugé. Au fond si nous adoptons si vous adopter ce projet de loi si vous votez. Le projet de loi de finances qui prévoira des crédits d'impôt industrie verte particulier qui sont une avancée majeure de la Commission européenne suscitée par la France. On sera à peu près au niveau avec les Américains. On a aujourd'hui quand on prend France 2030 quand on prend les montants autorisés par la Commission. Quand on prend les dispositions du dispositif temporaire lié à la guerre en Ukraine et quand on prend la possibilité de faire des crédits d'impôts dont la France se saisit dans le cadre de cette cette stratégie. On est à peu près au même niveau en termes d'encours. La réalité c'est qu'on a des approches philosophiquement différente que les États-Unis, ça va vite et très vite et donc il faut qu'on aille vite et très vite. Moi j'ai discuté avec le gouverneur de l'Idaho. La semaine dernière ils sont capables de donner une autorisation d'usine en 90 jours on ira pas jusque-là parce qu'on a des exigences environnementales auxquelles nous adhérons qui sont plus exigeantes dans 90 jours on n'y arrivera pas mais au moins, faisons en sorte qu'on aille à six mois on parallélisme les procédures. On ne met en aucun cas les. Les les enquêtes environnementales mais on va plus vite parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui donc l'Avantage compétitif de la France. Il est clair, c'est donc vous en déplaise, de l'énergie en grande partie nucléaire d'ailleurs décarboné pas cher et en volume. Ça, ça attire les investisseurs internationaux. Sur les montants, on est à peu près au même niveau sur les procédures, il faut qu'on aille plus vite et c'est vraiment l'objet de ce ce projet de loi dont je vous engage tous et toutes à le à le voter. Merci. Merci. Je mais on voit le 289 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Rejeté. On essaie de faire l'article 10 à l'article 10, le six Monsieur Salmon. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, l'article 10 prévoit de reconnaître à un projet la qualité d'opération répondant à un air 2 IPM dès la phase de déclaration d'utilité publique du projet. Le principe de regroupement d'autorisation et l'idée de mieux anticiper pour faire en sorte que les projets ne répondant pas aux droit de l'environnement et aux autres réglementations soit arrêté en amont et très utile. C'est mieux qu'à un stade avancé ou des dommages environnementaux aurait déjà pu avoir lieu. Bien entendu, cela peut également permettre d'accélérer les projets et à avoir une vision plus globale. Cependant ce dispositif pose plusieurs problèmes. Tout d'abord la reconnaissance de cette qualité ne pourra être contestée devant le juge administratif qu'au stade de la DUP et non plus au moment de la délivrance de la dérogation espèces protégées. La DUP a lieu tôt dans la procédure car l'expropriation prend du temps. Dans le cas où le projet concerné a des impacts sur l'environnement, le dossier comprend bien une étude d'impact, mais celle-ci, il faut le rappeler, n'est pas équivalente à une demande de dérogation espèces protégées qui comprend l'obligation d'analyser l'ensemble des espèces et les les espèces protégées. Bien entendu, espèce par espèce et s'assurer notamment avec les mesures éviter. Réduire compenser adéquate qu'il n'aient pas porter atteinte au bon état de conservation d'aucune de ces espèces protégées, déclaré que l'enveloppe des projets d'intérêts nationaux de trouverait pas être soustrait excusez-moi là, je suis passé sur l'autre feuille. Je m'arrête là. Merci. Avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. Chers collègues, l'amendement effectivement propose la suppression de l'Arctique lorsqu'elle est déclarée d'utilité publique d'un projet, il peut parfois se passer, vous le savez, de nombreuses années pour que le projet se concrétise et que soit demander si nécessaire une dérogation espèces protégées. Cette dernière peut être accordée. Mais vous le savez à 3 conditions cumulatives. D'abord la reconnaissance que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur je je vous connaissez les 2 autres conditions si ces deux dernières conditions justement ne peuvent s'apprécier qu'en fonction du site exacts retenus et de la forme finale du projet, son caractère R 2 IPM est appréciée dans l'absolu au regard des bénéfices pour la collectivité mis en balance avec les inconvénients par exemple de nature environnementale, mais sans perdre en compte spécifiquement à ce stade, la question des espèces protégées. le caractère 2 IPM peut donc s'apprécier bien en amont de la relation du projet si ce dernier est suffisamment avancée. L'Arctique propose uniquement d'avancer la reconnaissance R 2 IPM pour purger le délai contentieux avant la réalisation du projet mais la dérogation espèces protégées pourra toujours être refusé aux deux autres motifs. Ce sera donc un avis défavorable à cet amendement.

quand vous des des décidé qu'un qu'un projet d'intérêt national majeur là il nous a, au contraire, autorisés à mettre en cohérence de notions très proches dans la loi aujourd'hui qui peuvent apparaître. Incompatible donc l'utilité publique qui permet l'expropriation et la R IPM qui permet, dans certaines conditions le rapporteur de la merde il a des révélations aux histoires d'espèce protégée, donc on essaie de mettre en cohérence. Les deux aires IPM utilité publique c'est ce que l'article 10 permet de faire donc un avis défavorable à cette amende.

Oui, monsieur le Président, cet amendement de notre collègue Marta de Cidrac vise à recentrer le dispositif de l'article 10 sur les seuls projets industriels en cohérence avec l'objet du texte. Il semble en effet plus pertinente dans un texte consacré au projet d'industrie verte de ne pas ouvrir trop largement le bénéfice du nouveau dispositif. Seule la déclaration d'utilité publique des projets industriels pourraient ainsi le reconnaître le caractère d'opération répandant une raison impérative d'intérêt public majeur c'est ce que nous avions fait également dans la loi dans la

se on se tient on se cantonne à l'objet de ce projet de loi, on aurait tendance à comprendre à la logique de votre amendement mais ça risque de complexifier un peu l'histoire. On vous souhaite vraiment mettre en cohérence, ces 2 procédures je dirais pour l'ensemble des projets, même si certains d'entre eux évidemment ne sont pas industriel donc avis défavorable. Je mais aux voix le 69 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 10 qui est pour.

Vivre à étendre la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale à l'ensemble des EPCI en vue de favoriser le regroupement des surfaces de vente pour libérer du foncier économique à titre expérimental pour 3 ans. Merci avait la commission. que monsieur le président, Monsieur le Ministre. Pour rappel, le gouvernement a lui-même dans la loi 3DS prévu la possibilité d'expérimenter sur une procédure unique d'autorisation en matière d'urbanisme commercial ou l'autorisation d'urbanisme tiendrait lieu d'autorisation commerciale sans qu'intervienne la CDAC cette expérimentation dans le système de la loi 3DS n'est possible que dans le cas d'une opération de revitalisation des territoires, nous voulons, pour notre part, lever la contraint de la contractualisation avec l'État, car nous faisons confiance aux collectivités qui sont responsables et qui n'ont pas besoin donc d'être accompagnés. Je rappelle que les autres critères très instructif fixées par l'article 11 demeure dans tous les cas par Dati pas d'artificialisation nouvelle et pas de création de surface de vente supplémentaires, c'est donc un avis défavorable. Mais aux voix l'amendement 321 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est compte. Moi. Le 410 monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président, j'ai conscience que cet amendement a été déposé un un peu d'hardiment donc je tiens à vous en présenter nos excuses. Mais pour autant c'est un amendement important. Qui complète l'article 11 relatifs au transfert des autorisations d'exploitation commerciale dans la grande opération d'urbanisme pour rendre la goût plus accessible et efficace. Il s'agit d'un appel d'un amendement pardon d'apparence technique très important. Que la ministre ma collègue en charge des PME du commerce et de l'artisanat Olivia Grégoire construit depuis 8 mois, avec les parlementaires, je pense. Certains d'entre vous en tout cas les élus locaux en lien avec le Conseil national du commerce. Il propose de compléter l'article 11 qui prévoit comme vous le savez d'exonérer une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale. Les opérations de remembrement commercial s'inscrivant dans les grandes opérations d'urbanisme. C'est-à-dire concrètement, accélérer la transformation de zones commerciales dont on sait qu'elles font face. À des défis énormes liés à la transformation des modes de consommation de nos concitoyens pour qu'elles puissent accueillir de nouvelles activités comme de l'industrie. Je souhaite vraiment que cet amendement soit puisse être adopté et suis impatient d'entendre et de ce fait l'avis du rapporteur. on va lui demander son avis. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre sur le. Principe desserrer les contraintes qui pèsent sur les collectivités en matière d'aménagement et d'urbanisme uniquement dans le cadre de partenariat que l'État nous gêne un petit peu. En outre, la méthode qui consiste à proposer dans un projet de loi une mesure intéressante et en restreignant le périmètre de sorte à la rendre inopérante pour faire passer une réforme du régime du régime de ce périmètre est aussi assez curieuse mais enfin bon. Une telle réforme aurait mérité sûrement davantage de concertation, je reconnais cependant que cette réforme lève une importante restriction de la goût auquel était très défavorable. Madame la présidente de la commission des affaires économiques qui a manifestement freiner son acceptation par les communes, à savoir l'obligation de transférer la compétence de délivrance des autorisations d'urbanisme à l'établissement public de coopération intercommunale. Ce sera donc un avis de sagesse. Monsieur manteaux. Non. Le retrait. Très bien je vais donc mettre aux voix cet amendement du gouvernement avec un avis de sagesse. De la commune. Sion, qui est pour. Qui est contre. Cet amendement est adopté. Je je mais aux voix l'article 11 ainsi maudit. Qui est qui Qui est contre. Il est adopté. La présidente on finissait là l'aspect économique avec les quatre ou cinq amendements après l'article 11 comme vous voulez. Soit on termine, comme ça on fait le bloc écho. Soit soit vous avez un problème et on enlève. Monsieur le Ministre. Très bien, donc après l'article 11, le 160, Monsieur Montaugé. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc le le ministre de l'Économie et des Finances nous a indiqué à l'audition. Qu'il voulait garantir la la délivrance des autorisations nécessaires à un porteur de projet industrie verte dans un délai de 9 mois. Cette ambition suppose une coordination et une organisation adaptée des services de l'État. Pour assurer la bonne application de la loi, l'efficacité et la lisibilité de l'action de l'État. Nous proposons. Avec cet amendement, que le gouvernement prenne un décret pour définir les modalités qui permettraient d'assurer la mise en oeuvre des mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches et les moyens qu'il entend affectée à ce chantier

Cette mesure proposée va dans le sens d'un meilleur suivi de l'application de la loi que nous promouvons, ça ça donnera plus de visibilité à quoi ce suivi. C'est donc un avis favorable. Monsieur le Ministre, allez même avis Mets aux voix l'amendement 160 avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Toujours après l'article 11 4 amendements identiques. Le 152, Monsieur Montaugé. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le le développement industriel dans les territoires pourrait davantage s'appuyer sur le programme territoires d'industrie et sur les acquis méthodologiques de la première phase du dispositif donc intitulé territoires d'industrie. Territoires d'industrie est un instrument efficace. Moi je le constate sur mon territoire. En tout cas une partie de mon territoire et et. Outil de reconquête industrielle, il est perçu par les élus locaux et les chefs d'entreprises industriels comme un cadre important de dialogue et de soutien aux projets territoriaux. Il était indispensable car la politique industrielle reste reste encore bien trop concentré au plan territorial. Plus de 40% des aides à l'innovation par exemple sont fléchés sur seulement 5 départements français. Une nouvelle phase du programme sur 2023 2027 donc territoires d'industrie a été annoncée par le président de la République et-ce plutôt une, une bonne nouvelle. Avec cette demande d'appel Monsieur le Ministre, nous souhaiterions connaître le bilan actuel de territoires d'industrie. Et les intentions du gouvernement sur le périmètre de la nouvelle génération du programme territoires d'industrie les les entreprises. Partie prenante des des chaînes de valeur concernant les, les grands sites industriels objet du, du projet de loi industrie verte il auront telle accès.

Oui, monsieur le Président c'est un amendement identique à un amendement d'appel relatif aux territoires d'industrie. Si le 257 monsieur

Comme tous nos collègues, monsieur le président. Et nous sommes attachés au programme territoires d'industrie lancée en 2018 qui concerne actuellement 150 intercommunalité ou groupes d'intercommunalité City situé en zone rurale, particulièrement dans les espaces péri-urbain, les petites villes, petites ou moyennes qui présente une forte identité un savoir-faire industriel les plans d'action élaboré dans le cadre du programme vise notamment à renforcer l'attractivité des territoires pour le développement entre autres via un soutien au recyclage foncier et à la revitalisation des friches industrielles à la fourniture d'd'ingénierie, des projets et le développement des écosystèmes locaux industriels cet accompagnement ciblé plébiscite plébiscité par les acteurs locaux il rentre parfaitement je dirais dans cette loi industrie verte il semblerait tout à fait pertinent de faire bénéficier davantage de territoires de ce dispositif. Pour cette raison monsieur le président, ce sera un avis favorable pour les amendements. 152 181 257 372 et 334 si les rectifier pour être identiques aux 3 autres. À dévorer la Bible qui est le le le dossier de presse du, du projet de loi industrie verte dans lequel un certain nombre. D'éléments précis avait été avait été précisé. C'est un programme exceptionnel. C'est un programme, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs qui permet d'aligner tout le monde. De mettre en place dans un territoire mais il faut le reconnaître, plutôt dans les territoires éloignés, dans les territoires ruraux dans les territoires. Périurbains dans lequel l'industrie a été importante et ne l'est plus, ou dans lequel l'industrie recommence à être importante et on souhaite l'accompagner et moi je préférerais qu'on se focalise sur ces territoires-là les territoires que vous mentionnez dans votre abonnement franchement ils vont bénéficier des projets d'intérêt national. Ils vont bénéficier d'un certain nombre de dispositions de cette. De cette loi. Donc moi j'engagerai vraiment plutôt à retirer ses amendements mais retenez quand même que ce qu'on fait en territoire d'industrie c'est 100 millions, à condition tout ça évidemment soit votée dans le cas des projets de loi de finances à venir une enveloppe budgétaire annuelle de 100 millions pour appuyer les investissements industriels dans les territoires actualiser la carte des territoires d'industrie parce que certains qu'il était non peut-être plus beau caution à être mais au contraire certains qui n'était pas encore quand on a lancé le programme pourrait le devenir. Et surtout il y a un certain nombre de dispositions. Une disposition extrêmement importante pour moi mais je pense aussi pour vous, c'est le dispositif rebond industriel qui permet d'accompagner des territoires qui aujourd'hui font face à des difficultés extrêmement importante de manière à les accompagner vers l'avenir. Ce dispositif a été extrêmement utile dans le territoire de Béthune suite à la fermeture de Bridgestone et il est aujourd'hui lancée dans le territoire de Caudry dans lequel vous savez qu'on a un défi. La fermeture programmée pour lequel nous cherchons et nous espérons encore trouver un repreneur de l'usine dite de Buitoni et la fermeture programmée de la sucrerie de Téréos pour laquelle nous travaillons, je peux vous dire avec un peu de pression, d'ailleurs sur l'entreprise pour qu'elle puisse. Aller gérer au mieux cette fermeture et ce programme il est vraiment extrêmement utile, il est dans le cas de territoires d'industrie il va être maintenu, donc je vous engage et merci de ce soutien à continuer à soutenir ce ce ah les disette budgétaire difficultés budgétaires sur les territoires qui en ont le plus besoin donc demande de retrait. Bien. Madame Paoli-Gagin est-ce que vous. Modifiez votre amendement pour le rendre identiques aux autres.

je n'ai jamais compris et je et, je l'ai dit. À de multiples reprises. Pourquoi on ne se focaliser. Sur la périphérie des métropoles et qu'on laissait des pans entiers du territoire sur lesquels on avait des entreprises industrielles.

du du du du gouvernement ou des gouvernements. Incompréhensible quoi et et et pas très bien vécu. Voilà donc moi je me réjouis qu'il ait pu ce critère finalement en tout cas si je l'ai bien compris le le le le la nouvelle étape qui est plus ce critère de de localisation géographique. Parce que c'est fondamental et et c'est surtout dans l'intérêt général national. Que d'embarquer. Dans en matière industrielle lance un de territoire, y compris les territoires ruraux souvent agricoles ou 13 agricole qui rend compte par ailleurs des difficultés le développement industriel, c'est aussi un moyen de relancer le développement de ces territoires parfois hein hein. Difficulté. et merci je je tiens à le dire en même temps. Merci à la DGE et à l'équipe de Monsieur Gueusquin qui travaille de manière remarquable sur ce sujet et qui sont vraiment dans l'écoute des territoires et des élus locaux que nous sommes. Très bien. Madame variable. de relocaliser réindustrialiser notre pays c'est une démarche évidemment que l'on peut soutenir mais dans le même temps. Effectivement, il me paraît essentiel de préserver aussi nos savoir-faire. Et aujourd'hui, et j'en veux pour preuve le couperet qui viennent de tomber dans mon département en Dordogne sur les papeteries de Condat-le Lardin. Qui sont qui la seule entreprise en France à détenir le savoir faire de la fabrication du papier couché double-face dans le groupe. L'État a transféré cette chaîne. En Espagne. Bien sûr, pour produire à moindre coût aujourd'hui sur 420 salariés, 187 suppressions de postes, 2000 emplois induits dans l'économie dans notre ruralité. Donc effectivement je pense que. Si la démarche est louable de réindustrialiser. Je crois qu'il faut accompagner ce savoir-faire nous avons il y a un marché, il y a un marché sur ce papier couché je pense aux, aux élèves, aux éditions Gallimard, Flammarion, Hachette et cetera. Nous avons le devoir et je sais, Monsieur le Ministre et je remercie votre cabinet d'avoir répondu à ma demande de de d'd'entretien je je m'en félicite mais je pense que là nous avons une bataille à mener, en tout cas je serai aux côtés des élus et nous la mènerons jusqu'au bout parce qu'il est inadmissible que nous ne puissions pas. Alors que dans le même temps, ils ont installé une chaudière biomasse qui a été très largement. Subventionné par l'État, la région à plusieurs reprises. Très bien. Monsieur le Ministre. Si Monsieur le Président. D'abord pour le sénateur Montaugé alors le programme territoires d'industrie c'est pas un bar ouvert pour tous les territoires. Il y a vraiment une condition de mobilisation très forte des élus locaux et de l'écosystème pour porter un territoire vers l'industrie et donc c'est vrai que dans la première fournée de territoires d'industrie et j'allais dire dans la 2ème. Ce sera la même chose, on a besoin d'avoir des projets dans quel ensemble tout le monde est motivés, mobilisés pour accompagner et je dirais c'est du donnant, donnant, si vous êtes prêt, nous sommes prêts, vous l'avez dit, les services de l'État sont exceptionnels et donc merci des bons mots que vous avez eu à leur égard. Mais on est quand même dans une démarche de labellisation les, les fonds sont limitées, on souhaite les concentré et évidemment le Gers et tout à fait aussi. Autorisés que les autres départements a. À postuler à ce Label. Et si les projets sont au rendez-vous. Mais il y a aucune raison que le Label territoires d'industrie ne soit pas non plus lui au rendez-vous Je dirais. Conforté réconforté accompagner des projets qui sont déjà dans une dynamique locale évidemment si vous connaissez les services. Vous êtes prêts à leur présenter. De manière précise un certain nombre de de dossiers dans notre territoire concernant la la papeterie dossier que vous mentionnez, madame la sénatrice, vous le savez, il y a deux lignes dans cette papeterie. Une ligne qui fait du carton qui est extrêmement moderne qui a été accompagné par l'état d'ailleurs et la région et qui va continuer. Une autre ligne, vous l'avez dit qui fait du papier plus traditionnel dans lequel l'outil de travail et malheureusement. Très ancien. Obsolète moi ce qu'on dit c'est qu'il faudrait 80 millions d'euros pour investir dans cette nouvelle ligne de production. Alors que d'autres lignes similaire et compétitive existe ailleurs. L'entreprise a décidé du coup de délocaliser cette ligne de production s'est engagée auprès de nous, à maintenir la première. Nous allons évidemment nous assurer, vous l'avez dit, les services de l'État sont déjà à la manoeuvre que l'entreprise que la pérennité de l'entreprise est assurée avec une seule ligne de production plutôt que de qu'évidemment le plan de sauvegarde de l'emploi qui concernera sans doute une partie des employés il à la fermeture de la 2ème ligne sera je dirais au rendez vous des conditions sociales nécessaires pour les salariés.

Qui est contre. Ils sont adoptés. Je vais suspendre la séance elle sera reprise à 14h 45 pour la nouvelle lecture de la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatif. La séance. Est suspendu.